La séance est reprise, nous allons reprendre la discussion du PLF mais la parole est à monsieur bonhomme pour une mise au point sur un vote qui la parole. Oui, merci Monsieur le Président, oui effectivement je souhaite faire la mise au point suivante sur le scrutin numéro 67 pour vous indiquer que mon collègue Jean-Raymond Hugonet sauter voter pour. acte et donner votre mise au point, sera publié au JO, il figurera dans les risques politiques du scrutin nous reprenons donc la discussion du projet de loi de finances

Monsieur le prison, monsieur le rapporteur, messieurs les Ministres, chers collègues, l'examen de la mission fonction et transformation publiques me permis d'interpeller le gouvernement sur les affectations en général des fonctionnaires dans ma collectivité d'outre-mer, ne me dites pas que je suis hors sujet parce que les affectations en Outre-Mer d'expatriés ont un coût non négligeable pour le budget de l'est pas, en effet, Monsieur le Ministre, pour l'ensemble des différents départements ministériels concernés, celui de la justice et de l'Intérieur mérite votre attention au vu de notre actualité locale, comment peut-on encore aujourd'hui favoriser l'affectation d'un expatrié au détriment d'un Polynésien à compétences égales,

que des originaires de Polynésie et en exercice dans l'hexagone depuis plusieurs années, attendez leur mutation, un collectif a été emporté par le ministre Darmanin que je remercie par ailleurs, je m'interroge aussi sur le choix de certains candidats métropolitains affectés chez nous, on entend, on découvre des comportements des propos sévères dans l'exercice de la fonction à l'égard du personnel polynésien et c'est le cas à d'action de la police nationale de propriété, je mets interroge fortement sur ces mouvements de personnel ainsi, Monsieur le Ministre, de grâce, veiller à plus de vigilance dans le choix des affectations en outre-mer et veuillez donner instruction aux administrations centrales pour un meilleur respect des dispositions de la loi élan et les critères de du C. car il y a un réel sentiment de malaise qui se développe une rencontre parmi nos fonctionnaires polynésien, une perte de confiance à l'égard de l'État avec ces affectations dans le coup, est important pour le budget de l'État avec des avantages financiers se rattachant à l'expatriation, monsieur le Ministre, ces affectations dictée de Paris font beaucoup de mal, chez nous, on le ressent de plus en plus je conclus Monsieur le Président, et il ne faudra donc pas s'étonner que les non indépendantistes progresse dans les mois à venir, je vous remercie.

Merci beaucoup monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des lois sur le président de la commission des des finances je tiens aussi à saluer le travail des rapporteurs spéciaux Claude nous Mougin Albéric de Montgolfier, Sylvie Vermeillet, ainsi que les rapporteurs, Paul Paul Paul René Savary et Catherine Di Folco pour tout le travail qui a été réalisé, je dirais concernant j'irai cette mission, mission importante qui regroupe, je dirais à la tronche, transformation, fonction publique, gestion du Patrimoine immobilier de l'État, mission de gestion des finances publiques régimes sociaux, retraites, pensions, donc c'est vraiment je dirais très très important comme engagement financier, donc, pour le temps qui m'est imparti je j'aurais aussi comme d'autres collègues qui se sont exprimés, hein, un manque de respect pour le l'inspecteur de des finances publiques qui a perdu la vie dans des circonstances dramatiques lors d'un contrôle fiscal dans le département du Pas-de-Calais puis également on insouciant, la douleur de la famille des proches et aussi bien entendu de ses collègues, parce que je crois que c'est aussi des Liens importants de solidarité que nous devons avoir les marques de respect et de reconnaissance pour l'ensemble des fonctionnaires, je dirais que ce soit la fonction publique d'état fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière et se

des femmes et des hommes, je dirais qu'ils sont au service de nos concitoyens, des habitants et puis qui se dévouent beaucoup 5 66 millions d'agents qui sont répartis pour la fonction publique d'État, soit 45 % des effectifs pour la fonction publique territoriale 34 % à la fonction publique hospitalière 21 % et dans le projet de loi de finances pour 2023 est prévue normalement la création de plus de 10000 emplois équivalents tremplin notamment donc plusieurs ministères Éducation nationale Justice intérieur et je voudrais je voudrais évoquer aussi principalement je dirais m'attarder un petit peu sur la la la gestion des des finances publiques, notamment la direction les directions DGFIP auquel nous sommes attachés à l'échelon du départ de nos départements et territoires respectifs puisque je dirais malheureusement depuis pas mal d'années, les effectifs ont été réduits en moyens humains certes

peut être dans certains cas, efficace, mais c'est aussi des personnes qui sont les, les, les trésoreries était au service aussi de son service de nos collègues élus l'ordonnateur et elle comptable et c'est vrai que c'est réellement important cette présence humaine, auxquelles nous sommes attachés, puis également, ils sont aussi à l'écoute de nos et et le et également les particuliers, avec aussi des, des, des, des missions qui sont réellement très importantes j'associerai aussi à mes propos, l'administration des est du ressort de l'école du ministère de l'Économie et des Finances, puisque je représente les Ardennes, département frontalier dans lequel les douanes joue aussi un rôle très important aux côtés de nos forces de sécurité intérieure et à ce niveau-là, je citerai le travail et celui où elle travaille aussi de nos collègues, Albéric de Montgolfier Claude Mougin sur un rapport intéressant qui était présenté en commission des finances récemment la douane face au trafic des des stupéfiants avec 11 recommandations et c'est aussi très important puisque nos collègues ont ont ont mesurer aussi l'engagement de l'administration des douanes, mais aussi les moyens qu'il convient de le reporter moyens humains bien entendu mais aussi moyens techniques sous toutes les formes, et je crois que c'est aussi très important voilà je conclurai en en saluant vraiment tout ce travail et naturellement Monsieur sur et on aux avis des des différents rapporteur pour soutenir ses différentes missions, je vous remercie. Merci, cher collègue là. Maintenant au ministre Stanislas Guérini le gouvernement dans son ensemble à dix minutes Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le, le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les sénateurs, d'abord merci pour vos mots sur tous les bancs, à à l'égard de cet agent du du service public, a perdu la vie en faisant sa mission en faisant son service et c'est bien l'argent, l'ensemble des agents de la fonction publique, vous avez raison de le rappeler qui sont aujourd'hui en deuil, je suis heureux ce soir d'être avec vous de pouvoir vous présenter le budget du ministère de la transformation et de la fonction publique, qui êtes en hausse de 57,8 millions d'euros quand on prend l'ensemble de ses missions, ce n'est pas le budget le plus important en volume que vous ayez à examiner, mais vous le savez très bien, c'est un budget de 2 leviers ai d'action qui permet d'enclencher un certain nombre d'actions pour la fonction publique, je reprendrai ici peut-être quelques faits saillants d'évolution des crédits budgétaires d'abord renforcer les compétences au sein de la fonction publique, c'est une des priorités, les uns et les autres avaient mentionné cette priorité autour de l'attractivité de la fonction publique, donc je ne mentionnerait le fait que nous ayons créé 7 emplois supplémentaires au sein de la direction générale de l'administration et les finances publiques pour porter justement, la réforme des carrières et des rémunérations qui sera un enjeu extrêmement important de l'année 2023 nous avons augmenté les moyens de la direction, hein, terminé, ça la transformation publique en créant 22 emplois justement pour renforcer nos compétences de conseil interne, c'est l'engagement que j'avais pris, ici au Sénat, comme nous avons eu à examiner la proposition de loi sur les cabinets de conseil, j'en profite pour dire aussi que l'autre engagement qui avait été pris qu'créer une annexe budgétaire dédiée un jaune budgétaire pérenne dans le budget a été tenue, puisque vous avez pu noter que ça fait partie des amendements qui ont été retenus et qui donc inscriront dans le temps dans le temps long cette annexe budgétaire importante je veux signaler aussi bien que ce ne soit pas stricto sensu dans ce budget, le renforcement considérable des moyens que nous donnons à la Direction interministérielle de l'encadrement supérieur de l'État la dièse, la DRH de l'encadrement supérieur de la fonction publique, c'est évidemment essentiel, est liée à la réforme de la haute font son public que nous conduisons et c'est-à-dire un objectif de transformation de l'action publique 2ème priorité qui se voit dans le budget rendent nos services publics plus efficaces et plus accessible, le choix qui a été fait, c'est de continuer d'investir dans la transformation de l'action publique en reconduisant le fond de transformation de l'action publique en consacrant transe 330 millions d'euros sur l'exercice 2023 2025 dont sur les 3 prochaines années et 120 millions d'euros dès 2023 moyens qui seront consacrés à des projets de transformation de l'action publique, bien sûr, vous l'avez mentionné aussi nous déployons encore et toujours les espaces France service en reconduisant les moyens pour accompagner les collectivités dans le déploiement des Maisons France service et en se dotant de moyens pour continuer à déployer 150 espace francs service supplémentaire sur l'année 2023 je veux à ce titre-salué la mesure qui a été portée par le sénateur Delcros dans le débat budgétaire qui a permis d'abonder encore de 12 5 millions d'euros, les crédits alloués à cette politique de service public, je dis aussi un mot sur le fait que nous pérennisons les moyens pour le développement des conseillers numériques France service ils nous aurons l'occasion d'y revenir, puisque un amendement porte sur ce programme là je veux enfin précisé que le gouvernement présentera un amendement visant à abonder de 2 millions d'euros, le programme 349 pour donner des moyens à nos services déconcentrés à nos préfectures pour porter les politiques prioritaires du gouvernement pour communiquer aussi sur les politiques prioritaires du gouvernement, je crois que c'est essentiel pour le suivi de nos politiques publiques pour la confiance de nos concitoyens envers l'action publique et puis je concluerai en disant un mot du financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale, vous l'avez mentionné tout à l'heure, madame la sénatrice d'abord en saluant effectivement un engageant maintenu pour l'exercice 2023 15 millions d'euros sur les crédits du ministère 15 millions d'euros via France compétences qui nous permettra de maintenir cet effort pour porter l'apprentissage dans la fonction publique, nous avions dépassé les objectifs 8000 apprentis objectif : dépasser avec 12000 apprentis sur l'exercice précédent, et ça nous donnera l'occasion d'avoir une discussion sereine avec le Cnfpt, avec l'ensemble des acteurs de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale pour trouver les bonnes conditions de financement de cette politique prioritaire, voilà les faits saillants que je voulais porter devant vous mesdames et messieurs les sénateurs et je passe la parole à mon collègue Gabriel Attal. Merci monsieur le président, messieurs les rapporteurs spéciaux, mesdames, messieurs les rapporteurs pour avis, monsieur le président de la commission des finances, mesdames et messieurs les sénateurs, le contexte d'incertitude auquel nous devons faire face nous invite à adapter en permanence l'action que nous conduisons je m'appuierai sur 2 exemples cités dans le cours de notre discussion sur le programme 348 nous mettons tout en oeuvre pour rattraper le retard pris par certains travaux depuis la crise sanitaire comme cela a pu être souligné depuis le début de l'année 2022 20 marché ont été notifiés l'ensemble des cités seront en chantier entre la fin 2022, et le début de l'année 2023 et les livraisons interviendront entre 2023 2024, ce programme a su s'adapter au contexte d'inflation, issus notamment de la guerre en Ukraine une priorisation a été opéré au sein des opérations planifiées afin de maintenir l'enveloppe fermée d'un milliard d'euros malgré l'évolution du coût des matières premières pour 2023 le programme 348 portera une nouvelle action résilience, d'un montant de 150 millions d'euros destinés à engager des travaux qui permettront rapidement de diminuer la facture énergétique des bâtiments publics sur le programme 552 dépenses accidentelles et imprévisible, nous avons provisionné 770 millions d'euros pour faire face aux conséquences de la crise énergétique et au contexte macro-économique monsieur nous Jean s'est étonné du montant de cette dotation, nous aurons eu nous aurons l'occasion d'y revenir au moment des amendements, nous pensons toutefois que l'État doit être extrêmement prévoyant et ne peut prendre le risque de laisser les Français démunis dans le contexte de crises à répétition que nous traversons, ces crédits pourront bien sûr être annulée en fin d'exercice, ils n'ont pas été utilisées malgré ce contexte d'incertitude, les directions de à la mission Gestion des finances publiques continuent de mettre en oeuvre des réformes ambitieuses, porteuses d'efficacité en matière de services rendus et de contribution à la maîtrise des dépenses, si les marges restantes sont moins importantes sur les emplois après les grandes réformes engagées par la DGFIP, tels que le prélèvement à la source, la suppression de la taxe d'habitation et la dématérialisation d'un certain nombre de profs et de le ministère poursuit ses efforts et notamment la DGFIP, avec 850 suppressions d'emplois en 2023 cette bonne gestion de nos crédits n'a pas pour effet de diminuer la qualité du service, la réorganisation territoriale de la DGFIP lui permet d'être désormais bien présente à moins de 30 minutes de 98 % des Français au sein du réseau des maisons France service parallèlement la direction et la direction générale des douanes poursuivent les réformes engagées de transfert des missions fiscales au global, les moyens supplémentaires qui sont déployées au travers ce PLF ont vocation à financer des priorités précisément identifiés, je pense à la modernisation de nos systèmes d'information, les augmentations relevés par les rapporteurs sur les crédits or titre de ont pour principal objectif de relancer une dynamique d'investissement et d'innovation forte au sein du ministère, je citerai notamment 450 millions d'euros annuels alloués à la modernisation des systèmes d'information, de la DGFIP, l'augmentation des crédits informatiques a vocation à résorber ce qu'on appelle la dette technique de nos systèmes d'information mais aussi à gagner en efficience, par exemple, pour répondre à la à l'intervention du sénateur Laménie sur l'organisation des moyens de la douane sur la lutte contre les stupéfiants, l'utilisation de ciblage issus du du Data Mining a d'ores et déjà permis de faire de la détection non intrusive de stupéfiants, la direction de l'immobilier de l'État pour sa part met en oeuvre une politique de rationalisation du Patrimoine bâti, afin de limiter l'empreinte carbone de l'État et prendre en compte le développement de nouveaux modes de travail, tels que le télétravail ou le Flex office je précise au rapporteur, et comme les comme les rapporteurs long nous y ont invités là des lieux privilégiera désormais une politique de redynamisation des redevances de modernisation du Patrimoine existant et de recherche de solutions alternatives à la session pour les biens difficilement cessibles tels que les baux emphytéotiques enfin les moyens que nous proposons d'allouer en matière de personnel vise à la fois à réinternalisation des prestations autrefois réalisées en externe auprès de consultants privés et à renforcer certaines missions comme Tracfin ou la cyber sécurité enfin pour terminer sur la question des retraites, de nombreuses questions ont été posées de façon légitime, nous les aborderons dans le cadre plus général de la réforme que nous conduirons en début d'année prochaine, je vous remercie et je veux remercier les rapporteurs, les orateurs des groupes de leur travail d'analyse très poussées sur les crédits d'émission examiné ce jour, je souhaite que nos échanges, nous permettent de répondre à l'ensemble des questions qui sont posées sur ses différentes missions. Merci, monsieur le Ministre. Nous en venons donc à l'examen des crédits des missions des comptes spéciaux des articles rattachés et je rappelle que pour cette mission, enfin, cet ensemble de mission là nous avons jusqu'à 22 et nous avons quand même ces amendements plus une série de votes de d'articles de missions, donc il faut que soit chacun soit attentif, autant donc nous commençons par le, la mission transformation et fonction publique figurent les taper et nous commençons par un amendement du gouvernement qui a été annoncé par le ministre tout à l'heure. Oui, monsieur le Président, c'est un amendement que donc j'ai mentionné dans mon discours à la tribune, qui vise à allouer 2 millions d'euros supplémentaires à la direction inter-la transformation publique pour donner des moyens de pilotage à nos services déconcentrés, vous savez que c'est pas toujours les services qui dispose des plus forts moyen de pouvoir piloter, les politiques prioritaires du gouvernement, les objectifs que nous nous sommes fixés que nous affichons, d'ailleurs, dans le baromètre de l'action publique, sur le terrain, leur donner des moyens de pilotage d'animation territoriale de communication aussi, donc c'était un mesures de renforcement de notre capacité de pilotage de l'action publique et donc je vous invite à soutenir cet amendement de renforcement de nos crédits. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur.

parce que le ce, ce programme 349 il nous semble entièrement possible de financer ces mesures sur les crédits existants isolé ainsi cette enveloppe relève davantage GIC d'affichage de crédit parce que il y a une sous exécution chaque année de 30 à 40 alors on souhaiterait que tous ces Budgets plutôt transparent et le plus exact possible, ça ne peut pas être exact, mais quand même, quand chaque année, il y a 30 à 40 % d'écart avec cette demande de budget, c'est la seule raison pour laquelle l'avis est défavorable et non pas sur le fond de ce médecin. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Peut-être insister un instant sur le besoin de fléchage de crédit sur l'État déconcentrer, nous avons besoin de renforcer les moyens donnés à nos préfectures au niveau départemental pour mieux animer nos politiques publiques et les objectifs prioritaires que nous nous fixons sur le terrain, je crois que c'est vraiment une condition de transformation de l'action publique de pouvoir comme nous l'avons fait pendant la crise sanitaire, piloté par le terrain est ensuite remonté si je puis dire, dans la complexité administrative, je crois que ces moyens là ils seront consacrés spécifiquement je prends ici l'engagement devant la Haute Assemblée ah ce pilotage territorialisée au plus près de nos concitoyens et donc je me permets d'insister quelques instants dans l'argumentaire pour soutenir le renforcement de de ses moyens. Je soumets au Sénat, c'est là que l'amendement du gouvernement avec un avis défavorable sur la forme, a dit le rapporteur de la commission, quels sont ceux qui sont pour.

Monsieur le président, monsieur le ministre, il s'agit donc d'un amendement de ma collègue Martine Filleul et concerne le financement des conseillers numériques, alors que la fracture numérique touche plus de 13 millions de Français accentue les situations de détresse d'isolement et de précarité, le déploiement depuis 2020, des conseillers numériques France service a permis d'engager une première démarche inutile inédite pour renforcer l'inclusion numérique cependant cet amendement prévoit d'allouer une enveloppe de 100 millions d'euros pour maintenir le financement des conseillers numériques France service à un niveau satisfaisant en 2023 et ainsi pérenniser le dispositif, en effet, si le gouvernement a annoncé un nouveau financement de 44 millions supplémentaires dans le PLF pour 2023 cette enveloppe correspond en réalité une baisse drastique de la subvention allouée au dispositif, alors même que la subvention actuelle ne couvre en moyenne que 50 à 75 % du coût réel des conseillers numériques France service donc c'est pourquoi plusieurs opérateurs finançant les conseillers numériques France service demande à ce qu'un financement minimal de 25000 euros par an et par poste soit couvert sur les 3 prochaines années, d'où l'objet de notre amendement, je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président, l'avis est défavorable sur cet amendement qui vise à majorer donc 200 millions d'euros, les crédits alloués conseil numérique dans le cas du du plan de relance 4000 conseillers numérique France service ont été installés et nous sommes d'accord avec vous, chers collègues, que que il joue un rôle essentiel sur nos territoires, toutefois, les crédits alloués en 2023 nous paraissent suffisants en effet si était plus élevés, les années précédentes, c'était en cas de lancement du dispositif et il faut également bien rappelé le mode de fonctionnement de ses conseillers, ce ne sont pas des employées du ministère, l'État finance leur formation et une partie de leur rémunération, mais le reliquat est assurée par l'employeur, c'est-à-dire une collectivité territoriale, une association, donc je pense qu'il faut y aller progressivement et donc c'est un avis défavorable. Le ministre. Oui, monsieur le président, je dirais, une demande de retrait ou sinon un un avis défavorable, pourquoi d'abord merci pour vos mots de soutien à l'égard de cette politique publique que nous sommes en train de construire et quand je dis nous, c'est les collectivités territoriales, le monde associatif, celui de l'inclusion numérique et l'État, tous ensemble, de lutte contre la fracture numérique, vous l'avez mentionné à la tribune, madame la sénatrice, c'est une politique publique absolument nécessaire aujourd'hui les 3 quarts des relations entre les Français et leur administration se font via le numérique, donc on a besoin de continuer à numériser mais l'autre chiffre important, c'est que 13 millions de nos concitoyens sont du mauvais côté de la barrière de la fracture numérique et sont durablement éloignés, ainsi, de nos services publics, donc on a besoin d'aller les former, d'aller les accompagner, de développer et les conseillers énumérer les 4000 conseillers numériques qui ont été déployés sur le terrain depuis 2 ans maintenant, avec les fonds du plan de relance, mène un travail absolument essentielle, là où je voudrais vous convainc couteau de retirer votre amendement, c'est que nous avons effectivement réallouer 44 millions d'euros sur les lignes budgétaires mais nous avons aussi emmener un reliquat de 28 millions d'euros issus du plan de relance, ça nous donne 75 millions d'euros en réalité pour financer cette politique publique et donc j'en profite ici pour dire aux collectivités territoriales qu'elles peuvent continuer à pérenniser ces emplois, nous garantirons le financement de tous les emplois qui sont renouvellement de court terme et puis sur ceux qui arriveront renouvellement ultérieur, nous continuerons à maintenir un haut niveau de financement à 100 % pour certaines collectivités 75 % pour une minorité des emplois y compris en 2023, l'État continuera d'être extrêmement engagé dans le programme conseiller numérique France service que je porte avec mon collègue Jean-Noël Barrot, c'est évidemment une priorité et nous sommes assurés d'avoir les fonds nécessaires pour porter cette politique publique. Madame l'Afrique

Abstention : il n'est pas adopté et nous passons à l'amendement défendu par Monsieur Sautarel. Houllier et soutenu par de nombreux sénateurs vise à financer l'équipement et l'accompagnement des élus en situation de handicap dans l'exercice de leurs fonctions, l'exercice d'un mandat local, hein, qui implique des gages de présence de participation d'investissements que certains élus porteurs de handicaps ne sont pas en mesure d'honorer, sauf à avoir bénéficié d'aides nécessaires aménagements particuliers matériel recours à des aides humaines ces aides ont un coût non négligeable qu'il est parfois difficile d'assumer aussi afin d'un assume aux personnes en situation de handicap, un accès réel aux fonctions électives, cet amendement souhaité par la PHP propose d'augmenter de 250000 euros, le budget du FI PHP FP afin de participer au financement de ses équipements,

qui est réduit à due concurrence, je vous remercie. L'avis de la commission du rapporteur. Merci monsieur le président, donc nous demandons le retrait de cet amendement qui vise à majorer les financements alloués au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, nous considérons en effet qu'il s'agit davantage d'un amendement d'appel pour un fond dans la logique de financement par les contributions des employeurs doit être préservé ses modalités de fonctionnement permet aujourd'hui au fond d'assurer ses missions avec de nombreuses conventions conclues avec les employeurs nous partageons bien sûr, les propos de nos collègues sur la nécessité de mieux valoriser insérer les personnes handicapées, la fonction publique le mise pourra d'ailleurs sans doute apporter quelques éclairages nécessaires sur les actions menées par le gouvernement dans ce domaine, c'est pour cela que, on fait une demande de retrait ou, à défaut des défavorable. Monsieur le Ministre. Oui, monsieur le président, exactement le même avis que monsieur le le le rapporteur, vous avez raison évidemment de soutenir la meilleure insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, j'ai eu l'occasion d'annoncer, la semaine dernière un certain nombre d'améliorations et d'avancée très importante en matière d'insertion des personnes ce genre de handicap meilleure reconnaissance des référents handicap lui mène une mission qui est absolument essentiel et donc on va maintenant reconnaître le rôle et la mission des référents handicap dans le référentiel des métiers de la fonction publique effort accru sur l'apprentissage pour atteindre les 6 % de personnes en situation de handicap apprentis dans la fonction publique, meilleur déploiement du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, elle fut Ph AFP, vous avez mentionné, mais le problème de l'amendement, vous portez ce qui porte sur l'insertion des élus et l'accompagnement des élus en situation de handicap, ce qui est pas l'objet du programme 148 qui vise à accompagner les agents de la fonction publique et donc je pour cette raison que je demanderais plutôt un retrait de cet amendement, mais dont je partage évidemment le fondement et l'objectif. Sur ce taré. Oui, merci Monsieur le Président, effectivement j'ai j'ai j'ai eu peur à vous entendre, monsieur le ministre et monsieur le rapporteur, que que qu'on ne parle pas des élus puisqu'effectivement on partage tous la bonne intégration dans la fonction publique territoriale et les actions qui sont conduites et les efforts qui sont faits par les uns et les autres pour accompagner les personnes en situation de handicap mais la le l'amendement que porte mon collègue et auquel bien sûr je je me joins à Philippe Houllier c'est la situation particulière des élus qui aujourd'hui sont pour ceux qui sont en situation de handicap, confronté à un certain nombre de frein pour exercer leur leur mandat, j'entends que le programme en question s'adresse effectivement au à la fonction publique et non pas aux élus, donc je, je, je, j'entends le la remarque de simplement je pense que sur le fond, c'est un sujet qui mérite que nous réfléchissions à à des solutions pour faciliter la vie démocratique et en tout cas l'engagement citoyen et et l'actif des élus en situation de handicap je ne vais pas le retirer, parce que c'est un amendement qui est porté par mon collègue mais mais j'entends les les remarques et et j'espère qu'au-delà du vote sur cet amendement et puis y avoir une réflexion qui s'ouvrent sur ce sujet, je vous remercie. Je mets aux voix l'amendement proposé par le collègue et qui a fait l'objet d'un avis demande de retrait de la part de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. L'abstention, il n'est pas adopté, nous allons maintenant passer le vote des crédits de la mission que j'ai annoncé tout à l'heure, transformation et fonction publique, je n'ai pas eu de demande d'explication de vote avant le les deux la limite et je rappelle que la commission des finances, est favorable à l'adoption des crédits de cette mission je mets aux voix les crédits de la mission qui est pour. pour. Abstention : ils sont adoptés. Nous procédons maintenant à l'examen de l'amendement portant sur les objectifs et indicateurs de performance de cette même mission transformation fonction publique figurant à l'étage et amendement présenté par Madame Di Folco au nom de la commission des lois. Merci monsieur le président, là j'en ai parlé dans le lors de la discussion générale et les deux indicateurs de performance relatifs à l'action sociale interministérielle qui figurait dans le programme annuel de performance du PLF 2021 ont été remplacés dans le PLF 22 et dans le PLF 23 par un indicateur de performance unique qui est le taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d'action sociale, je pense que cet indicateur n'est pas pertinent, d'une part, il ne permet pas de connaître le coût de gestion des prestations d'action sociale dont la maîtrise demeure un enjeu important et d'autre part, le taux de satisfaction des bénéficiaires atteint déjà un niveau très élevé, si bien que les marges de progression pour les années à venir sont très faibles, par ailleurs, à l'heure où l'État prévoit d'ouvrir 135 places supplémentaires en crèche pour les agents, la question du coût moyen de réservation d'une place en crèche, continue de se poser, c'est pourquoi le présent amendement vise à remplacer l'indicateur de faire performance taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d'action sociale par les 2 autres indicateurs qui étaient utilisés jusqu'à il a, il y a 2 ans encore, coût de gestion des prestations des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d'action sociale et coût moyen annuel de réservation d'une place en crèche, ce qui me permet, ce qui me paraît beaucoup plus pertinent, je vous remercie. L'avis de la commission monsieur rapporteur. Merci Monsieur le Président, c'est un avis de sagesse sur cet amendement, de Madame, la rapporteure pour avis de la commission des lois, les indicateurs proposés sont liés à des données dont nous ou vont disposer dans des documents budgétaires, cependant nous partageons son avis sur l'insuffisance du nouvel indicateur de performance relatifs à l'action sociale interministérielle doux satellite chaise sagesse. Plutôt une demande de retrait, monsieur le président, mais je, je ne suis pas loin de partager la la ville de sagesse, c'est pas un enjeu budgétaire stricto sensu, j'essaie, c'est plutôt de vous expliquer, qui a été la logique de la direction générale de l'administration de la fonction publique, d'abord vous apporter une réponse sur le fond et vous indiquer que l'indicateur coût de gestion a diminué de 5 recettes % entre 2000 19 et 2021 et l'indicateur du coût moyen annuel de réservation en crèche est passé de 8475 euros à 7402 euros dans la même période, donc on a considéré que ces 2 indicateurs, mettait en lumière des coûts de gestion raisonnable et plutôt non excessif et ce qu'dans le bon sens, ils ont été remplacés par un indicateur plutôt de performance, c'est-à-dire de satisfaction à l'égard des usagers qui sont les agents publics qui bénéficient de ces programmes d'action sociale, donc ça correspond plutôt à une volonté de simplification des indicateurs pour aller directement à la satisfaction de ceux qui en bénéficient, donc c'est la raison pour laquelle la direction générale de l'administration et de la fonction publique ah j'ai plus pertinent d'avoir cet indicateur unique qui était un pilotage par la performance, mais je n'en ferais pas une grande affaire, voilà ce que je voulais vous syndiquer. Madame Di Folco. justement j'ai j'ai pas du tout envie de le retirer, parce que moi, en tant que rapporteur, j'ai besoin des indicateurs chiffrés, plutôt que d'un taux de satisfaction parce que je pense que les agents ont plutôt sont plutôt satisfaits, effectivement, mais moi, pour mon rapport, j'ai besoin d'avoir des chiffres donc je maintiens, je maintiens Donc cet amendement fait l'objet dans la vie de sagesse, la commission des finances et du de la ville demande de retrait du ministre, quels sont ceux qui sont pour cet amendement 102. Y a-t-il des contre. Les abstentions, il y a donc adopté, nous pouvons maintenant de procéder au vote des crédits du compte spécial, gestion du Patrimoine immobilier de l'État, l'état des il n'y a pas eu de demande d'explication de vote sur ce sur ce compte spécial et je vous rappelle que la commission des finances, est favorable à l'adoption de ces crédits, je mets aux voix les crédits du compte spécial qu'elles sont ceux qui sont pour.

crédit sont adoptés, nous passons à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Gestion des finances publiques, toujours à l'. Les. Nous avons nos mon premier amendement de monsieur de lait, mais en l'absence de son signataire, ils tombent

Merci monsieur le président, c'est le ministre, comme évoqué dans la discussion générale, notre groupe souhaite renforcer les moyens du contrôle fiscal et pour compléter le propos de la discussion générale, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires vous diminuer donc les effectifs des agents chargés des contrôles, ce qui induit mécaniquement moins de contrôle et donc moins de redressement effectué avec des conséquences majeures: d'une part l'État perd des recettes, et au vu de votre vision franchement comptable, on ne peut comprendre comment vous pouviez refusé de maintenir même de créer des postes qui génère de manière significative des ressources supplémentaires, d'autre part, la fraude n'étant plus suffisamment combattu, elle devient financièrement, on peut dire rentable au vu et au su de tout le monde et ce n'est pas un bon message qu'on adresse là ou à nous citoyens. C'est un avis défavorable sur cet amendement, qui entend majorer les crédits alloués à la direction générale des finances publiques au seul but de créer des emplois supplémentaires, nous ne partageons pas cette vision d'ailleurs puisque il y a eu aussi un certain nombres de chiffre qui ont été données qui ne sont pas tout à fait exact ou plutôt ils sont exacts, mais un peu mélangé parce qu'il ne faut pas confondre au niveau du contrôle fiscal, les montants notifié et les montants recouvrer les montants notifié il peut mettre n'importe quel chiffre, ce qui est important, c'est ce qui rentre dans les caisses de l'État, or sur 2015 l'année qui est de référence pour votre démonstration, chers collègues, vous dites que, il y a eu 21 milliards sur la suite du contrôle fiscal, mais ces 21 milliards notifié. Et recouvrait c'était que 9 milliards 6. Et en 2021 les recouvrer ces 10 milliards donc il ne faut pas mélanger les recouvrer et le notifier et donc il a eu un milliard en plus, en 2021 qu'en 2015, ce qui prouve que le contrôle fiscal donc et beaucoup plus efficace pour les caisses de l'État qu'auparavant et s'il a moins de contrôleur fiscal aussi c'est que il y a eu des changements notamment le Data Mining qui permet sur les grosses entreprises et sur les gros recouvrement de contrôles fiscaux d'être beaucoup plus efficace que le contrôleur d'il y a 20 ans, 30 ans, qui allait contrôler le boulanger pour savoir s'il avait pris une baguette sans la payer. Monsieur le Ministre, quel est votre avis sur le moment. Oui, même avis que le rapporteur qui a beaucoup dit, on a au contraire des bons résultats du contrôle fiscal encore ces dernières années et on a des montants notifié et tout et recouvrer qui sont très importants qui sont en hausse, on le doit évidemment à l'engagement de nos agents, on le doit aussi au développement de nouvelles techniques dans le contrôle fiscal maintenant, notamment grâce à l'apport du numérique, on a près de 50 pour 100 des contrôles fiscaux, qui sont orientées guider via le numérique et via des algorithmes qui permettent notamment de cibler par exemple des entreprises. Qui semble plus plus sérieusement proche d'un d'une fraude que d'autres, voilà donc avis défavorable. Bien, alors j'ai une demande des explications de vote de Monsieur Bocquet, et ensuite une de Madame Goulet. Nous allons soutenir l'amendement de nos collègues écologistes parce que entendre dire le rapporteur, que vous voulez créer de l'emploi pour créer de l'emploi, non les moyens humains du contrôle sont indispensables numérique ne va pas tout régler d'ailleurs, pour l'anecdote, entre guillemets, si c'est une anecdote vous souvenez que le groupe l'entreprise Google, moteur de recherche mondialement connu, qui a son siège en Irlande, a été rattrapé par la patrouille y a quelques années, il devait 7 milliards d'euros au Fisc français et à l'issue d'une négociation avec Bercy, parce qu'on négocie son impôt dans ce monde là. Ils s'en sont sortis avec un milliard, mais si Monsieur le Ministre, un milliard, donc ils nous ont piqué 6 milliards, donc, le numérique va pas tout régler et en récompense pour Google, maintenant ils vont Google va aider l'État français a repéré les piscines non déclarés sur le territoire français, on est dans ce monde là, donc, le numérique, c'est qu'un outil, mais l'humain d'abord, pour contrôler les enquêteurs les vérificateurs les contrôleurs oui si on s'appuie pas là-dessus la DGFIP, je crois, a perdu 20000 emplois depuis 2000, donc moi je soutiens pleinement l'amendement de collègues écologistes. pour la fraude à la TVA et un certain nombre d'outils qui n'arrive pas encore à se mettre en route malgré, malgré les promesses, donc moi je crois qu'il faut plus de ressources humaines quitta évidemment les dispatchés dans différents services, on en a beaucoup, on en a sur les prix de transfert, on en a sur la coopération internationale, moi je voterai cet amendement dès demain. Bien Monsieur de salauds seulement monsieur le Ministre, sauf si vous voulez pas n'attendez.

dans la bonne voie, puisqu'on a un milliard de plus de de récupérer mais un milliard de plus, on peut faire encore beaucoup mieux, donc c'est avec aussi des des personnes qui y travaillent au quotidien avec des beaux outils des beaux outils numériques, bien entendu, mais on ne peut pas se passer de l'humain. Madame Prima, je rappelle qu'il nous reste 12 amendements qui reste trente minutes. Merci monsieur le président, j'ai juste une question à poser à Monsieur le Ministre, je voudrais savoir, sur 100 postes ouverts aujourd'hui sur cette fonction de contrôle combien sont vraiment ou vraiment des vraies personnes derrière et ce qu'il y a des postes qui sont non pourvus dans ces services là. Il pourrait pour des peut-être, aujourd'hui ou quand vous pourrez mais en tout cas je suis intéressé par ce chiffre-là. Monsieur le ministre, et ensuite on vote. On va vous trouver le chiffre évidemment vous le donner, enfin moi je, je, évidemment que le numérique ne veut pas remplacer du Mans et heureusement d'ailleurs. Et oui, il y a eu des réductions d'effectifs à la direction générale des finances publiques ces dernières années, c'est même je pense la direction qui a le plus contribué dans les réductions d'effectifs de l'état mon ministère, c'est, je crois, autour de 5 ou 6 % des effectifs publics c'était 85 % des suppressions de postes, ces 10 ou 15 dernières années, on sait ce que je veux dire c'est que l'essentiel des suppressions de postes n'ont pas été sur ces missions-là mais sur des missions de recouvrement qui ont été complètement transformées pour le coup par la porte du numérique, quand on fait le prélèvement à la source, quand on modernise avec les déclarations préremplies bah, objectivement, vous avez besoin de moins de monde pour gérer le recouvrement de l'impôt que quand vous aviez pas le numérique. Quand on supprime la taxe d'habitation, alors je dis un gros mot ici mais, objectivement, vous avez plusieurs milliers de postes qui était chargé du recouvrement la la redevance télé, qu'on supprime la je dis un gros mot sur certains bancs, il y avait aussi plusieurs milliers de postes qui était chargé de du recouvrement et de la collecte, donc je veux dire qu'il y ait des suppressions de postes, ça peut aussi signifier, c'est le cas en l'occurrence, qui est une modernisation, mais encore une fois sur le contrôle fiscal, on a vraiment pas à rougir de ce qui est fait aujourd'hui à Bercy cet été on a aligné Do un milliard un milliard trois qui nous ont payé mais grâce à nos agents non mais attendez, grâce à nos agents de la DV Annie qui ont enquêté pendant 10 ans, pendant 10 ans, il y a eu 10 ans d'enquête, par des agents d'une très grande qualité qui ont permis de mettre à jour ce qui se passait, donc voilà je j'insiste par ailleurs sur le fait que on est dans un contexte très contraint, que je ne lèverait pas le gage et que donc, si cet amendement est voté, les 150 millions d'euros sont prix sur des missions qui sont absolument essentielles pour le bien-être des agents, notamment sur les politiques RH. Et sur et sur le l'apport qu'il l'aurait fait dans leur travail, donc à vider doublement défavorable. Messieurs et ensuite, si vous voulez bien, on va voter puisqu'il reste beaucoup d'amendements sur lesquels on ne pourra pas débattre. Oui, d'accord, pardon, Monsieur le Président, mais on on. Faut quand même dire quelques mots. Il faut aller à la serpe tout le temps. Peut être que bientôt on viendra même plus et puis on adoptera les Budgets comme ça, non mais vous dites grâce au au travail des agents. Non, grâce au travail des lanceurs d'alerte. Mac Donald. Oui, oui, lanceurs d'alerte, d'ailleurs, qui sont toujours pas protégées et qui sont toujours plus mis en difficulté, a le secret des affaires. C'est une camarade de la CGT qu'à porter le fer sur cette question là, non, mais, mais, oui, oui, c'est public. C'est pas les agents et quand on vous dit qu'il a besoin de plus d'argent, parce que Madame Goulet a raison, les montages financiers sont toujours de plus en plus complexes. Et que pour un certain nombre d'agents, maintenant il faut des travail presque de vrais enquêteurs et il faut pousser les choses avaient des montages financiers dans plusieurs paradis fiscaux. Et quand vous dites on a augmenté. La remontée oui 2021 mieux que 2020, mais notamment, c'est sur les aides Covid qui ont été largement distribuées ben si, si, si, il y avait 7 milliards quatre on a recouvert 10 milliards 4 notamment, c'est des aides Covid qu'on a été recherché parce que beaucoup de sociétés ont été créées, et on a été en reprendre un peu, et heureusement. Mais autrement, au rock au sens je suis pas sûr qu'on gagne sur Word sur les 10 dernières années, et si on veut aller chercher les plus gros, les très grosses entreprises il y a besoin de plus de monde sur cette question là, parce que ces montages sont de plus en plus difficile et on le voit bien, plusieurs exemples ont été donnés, y compris avec des multinationales qui font des milliards de bénéfices sur notre territoire et qui paye aujourd'hui quasi pas d'impôts, et vous le savez, c'est une question d'ailleurs la taxation des GAFA nous en fait un combat pour l'instant on ne voit pas grand chose arriver. Nous allons voter sur l'amendement 109. Monsieur bonhomme. Merci monsieur Président très rapidement, moi je voudrais avoir quelques précisions par rapport au dispositif foncier innovant qui a été mise en place à titre expérimental qui a recours aux algorithmes pour savoir d'abord si vous avez fait une première évaluation de cette expérimentation, et si vous envisagez de de l'éteindre. Et quelles conséquences éventuellement, ça peut avoir ça en terme d'effectifs qui par ailleurs effectivement les les effectifs de contrôle, on le comprend, ne sont pas les plus attractifs continue parfois des pressions dans lesquels l'exercice se fait, quelles conséquences en tirez-vous donc par rapport à l'articulation avec ce dispositif innovant.

bien, monsieur le ministre. J'essaye de me restreindre dans l'expression parce que j'ai compris que, il y avait un temps contraint d'ailleurs il se il se passe quoi si on n'a pas fait tous les amendements avant la fin. On les reporte au week-end.

c'est nous, 500 millions de. Elle a remporté la première année, on sera, je crois à 700 800 millions l'an prochain, on est le 1er pays européen à avoir mis en place une taxe sur les GAFA et on est encore un des seuls à l'avoir fait, qui pousse au niveau européen, qui est moteur au niveau européen et au niveau international pour avoir une taxation minimale des entreprises justement pour éviter l'optimisation fiscale et les prix de transfert, c'est nous, on a même annoncé que l'année prochaine, on le ferait avec un groupe de pays européens en avance si on n'arrive pas à convaincre les autres, on est en première ligne dans la négociation à l'OCDE pour y parvenir, donc honnêtement sur ce sujet-là, je suis très à l'aise en vous disant qu'on est pionnier et moteur. Je mais aux voix l'amendement 109 messieurs et de ses collègues avec avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui pour.

Monsieur bah Paris un amendement 189 et la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, cet amendement est un amendement d'appel, il vise à confirmer la reconduction du protocole d'accord sur la transformation du réseau des buralistes telle que cela a été annoncé par le ministre des Comptes publics en effet au moment de l'adoption de la loi de finances pour 2018 en place la mise en place d'une trajectoire fiscale sur le tabac et en accord avec les impératifs de santé publique, ce réseau d'entrepreneurs indépendants, s'est engagé dans un projet de transformation du métier et des points de vente, l'objectif de ce plan de transformation et d'accompagner les buralistes dans la transformation de leur établissement et de leur activité commerciale afin de leur assurer un avenir moins dépendants du tabac et d'en faire de véritables commerçants d'utilité locale au service de leur territoire et de ses habitants avec 23500 buralistes répartis sur le territoire dont 44 % dans des communes de moins de 3500 habitants le buraliste incarne le commerçant de proximité par excellence, ce réseau en pleine transformation, s'était aussi rendu de plus en plus utile à son territoire et aux habitants, notamment en se faisant roller de service au public relais poste et vente de timbres encaissement de certains impôts, amendes et vente de billets de train et le présent amendement prélève donc 100 millions d'euros en autorisations d'engagement et 20 millions d'euros en crédits de paiement et pour assurer la pérennité, donner de la visibilité au réseau des buralistes, ce protocole d'accord et reconduit pour 5 années s'achèvera donc au 31 décembre 2027. Merci monsieur le président, dans nous demandant le retrait de cet amendement, nous comprenons bien entendu les inquiétudes de notre collègue alors que les buralistes ont dû faire profondément évoluer leurs activités ces dernières années, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a conduit l'État à leur confier la possibilité d'encaisser le paiement de certaines amendes ou redevance il faut enfin noter que pour 2023 65 millions d'euros de crédit sont ouverts pour le soutien au réseau des débitants de tabac, le protocole d'accord qu'on tienne tant des aides destinées à compenser par d'activité que des aides à la transformation de l'activité, le gouvernement prévoit de prochainement redéfinir les modalités de ces aides, ainsi que leur montant et leur répartition peut être ministre pour en dire plus, donc, demande de retrait sinon avis défavorable. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, et merci, monsieur le sénateur pour cet amendement d'appel qui nous permet de rappeler le rôle absolument essentiel des buralistes dans notre pays, c'est un rôle évidemment de l'Iran de lien social dans beaucoup de territoires c'est un rôle économique parce que quand vous avez un buraliste qui ouvrent quelque part ben souvent vous avez ensuite de l'activité commerciale qui ouvrent autour et malheureusement quand un buraliste ferme ben il peut y avoir des effets en cascade sur d'autres commerces, donc on doit être au rendez-vous pour soutenir nos buralistes, j'étais à leur congrès, il y a quelques semaines maintenant, j'ai encore échanger très récemment à Bercy avec leur président, Philippe Cohen, on travaille à un nouveau protocole j'ai donné une obligation de résultat pour les prochaines semaines, on a un peu de temps, puisque le protocole précédant s'arrête, mais vous savez que sur les aides à la transformation, et caetera, il nous reste quelques mois de décaissement donc il y a pas d'inquiétudes à avoir, on travaille au nouveau protocole il y a les fonds prévus dans le PLF 2023 pour accomplir la fin du protocole précédant et pour démarrer le suivant, on travaille de manière extrêmement étroite sur ce sujet là pour toujours mieux les accompagner, je précise qu'il y a un autre volet qui est pas un volet immédiatement financier de soutien aux buralistes, mais qui est extrêmement important, c'est le nouveau plan tabac que je présenterai aussi pour lutter contre les trafics et contre la contrebande de tabac qui est un véritable fléau. Et on a maintenant découvert en France sur notre sol des usines clandestines de cigarettes. On en a démantelé 2 récemment. C'est enfin, donc là on va monter encore en gamme, je peux vous dire sur les moyens techniques qu'on va mettre en place pour détecter et pour, je l'espère, aussi je négocie en ce moment avec mon collègue Dupond-Moretti pour renforcer les sanctions pénales de ceux qui font du trafic de cigarettes donc merci et demande de retrait puisque c'était un amendement d'appel. Pas Paris oui monsieur le président, Monsieur le Ministre, je l'avais indiqué, c'est à l'amendement d'appel, bien entendu, je vous remercie d'avoir appelé le rôle très important des buralistes comme commerçants de proximité et donc dans ces conditions, je retire mon amendement.

le Gaillac au en Ille-et-Vilaine, vous ne connaissez peut-être pas, mais ce sont quelques-unes des plus de 80 monnaie locale complémentaire qui existent aujourd'hui et pour pourtant 37 virgule 5 % de nos communes ont une monnaie locale qui circulent sur leur territoire, elle rassemble plus de 10000 entreprises, associations, l'objet de cet amendement est une mesure de bon sens, aider ce dispositif à se développer, ce dispositif qui fonctionne, qui aide à dynamiser les économies locales et accompagner la transition écologique des territoires ces monnaies locales ont un impact positif sur le territoire un paiement en monnaie locale génère entre 25 et 55 % de revenus supplémentaires pour le territoire qu'un paiement en euros, cet argent va donc profiter à l'économie locale aux entreprises à l'emploi, au pouvoir d'achats à faire vivre le territoire et les circuits courts, c'est pour cela que nous vous demandons d'investir dans un programme d'accompagnement au développement des monnaies locales à hauteur de 2 2 millions d'euros pour l'année 2023 pour changer de braquet parce que ces monnaies locales, ce ne sont pas, ce ne sont pas des gadgets sont un véritable outil au service du développement local, donc je compte sur vous, merci. défendu la avis de la commission sur ces deux amendements monsieur rapporteur. ce n'est pas le bon véhicule pour le développement des monnaies locales qui reverse certes une grande utilité au niveau local et ne nous semble pas qu'il revienne à l'État d'ouvrir des crédits pour ces actifs, même s'il peut bien sûr par le biais d'autres programmes territoriaux, les accompagner, il existe déjà aujourd'hui une cinquantaine de ces monnaies ce qui illustrent leur dynamisme et peuvent vivre leur vie seul. Le ministre. Donc je mets aux voix ces deux amendements ah non pardon je mets d'abord à l'amendement de Monsieur Bruillet, puisqu'il est différent, il est plus élevé, donc je mets au voilà monsieur monsieur brouillé avec double avis défavorable qui est pour.

alors même vote même vote de tout le monde il y a pas d'adopter, non plus, nous passons un amendement émanant de la commission des finances que peut présenter notre rapporteur. L'amendement présenté par Jean-François Husson, au nom de de la commission des finances, donc le présent amendement vise à financer par redéploiement de crédits, la première tranche de l'augmentation du nombre des officiers fiscaux judiciaires au sein du service d'enquêtes judiciaires des finances, il reprend la recommandation numéro 5 du rapport de la mission d'information de la commission des Finances relative à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui préconise de doubler d'ici 5 ans au maximum non, le nombre d'eau et lors de leurs travaux, les membres de la mission d'information, on peut constater que le nombre d'eau agit est très inférieur aux besoins réels du service alors que les magistrats se montrent unanimes sur l'expertise ce service dans les dossiers de fraude fiscale. Oui vous donner l'avis du gouvernement, monsieur le Ministre. donner les moyens pour les contrôles fiscaux et pour l'action de la DGFIP simplement pourquoi cet amendement est inopérant, parce qu'il prévoit des crédits supplémentaires en 2023 pour des officiers fiscaux judiciaires comme si tout d'un coup, il pouvait apparaître des nouveaux officiers fiscaux judiciaires l'an prochain, alors qu'il faut plusieurs années de formation qui y a des écoles pour ça. Et donc, en fait, vous pouvez ouvrir des crédits pour l'an prochain, les promotions, elles sont déjà en cours d'étude et donc les promotions qui sortiront l'an prochain, on sait déjà le nombre et donc il y a pas besoin de crédits supplémentaires puisqu'on a les crédits pour le nombre de nouveaux officiers qui arriveront à la DGFIP, donc avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Y a-t-il abstentions il est adopté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Gestion des finances publiques, sur laquelle il n'y a pas non plus : demande d'explications de vote dans un délai et je rappelle que la avis de la commission des finances, est favorable à l'adoption de des crédits de cette mission je mets aux voix, quels sont ceux qui sont peu. Quels sont ceux qui sont opposés. Ils sont donc adopté, nous passons à l'examen de l'amendement portant sur les objectifs et indicateurs de performance, de la même mission Gestion des finances publiques amendement présenté par le rapporteur général sur le 437. Créer un indicateur de performance au sein de la mission Gestion des finances publiques relatifs à l'efficacité des contrôles programmés par recours aux Data Mining, il reprend la recommandation numéro 2 de la mission d'information de la commission des Finances relative à la lutte contre la fraude et la l'évasion fiscale, la part des contrôles ciblés par l'Intelligence artificielle et Data Mining, qui est déjà renseignée dans le cas des projets et rapport annuel des performances ce jour-indicateur efficacité de la lutte contre la la fraude fiscale, alors que le gouvernement indique que le développement de ces nouvelles techniques d'analyse d'eau permet d'améliorer la programmation des contrôles et de détecter les cas de fraudes les plus graves et les plus sophistiqués, il est impératif que davantage d'informations soient transmises au Parlement sur l'efficacité réelle de cette ces technologies ainsi que sur les progrès accomplis. On parlait tout à l'heure du Data Mining, effectivement il progresse en les la part des contrôles fiscaux fiscaux des entreprises programmée sur la base de Data Mining, c'était 30 % en 2020 45 % en 2021 et on finira à 50 pour 100 en 2022 je précise. Que ça démarre par du Data Mining, mais il y a toujours de l'humain, évidemment qui feront en charge le dossier voilà et donc pourquoi cet amendement est inopérant bah parce qu'en fait c'est c'est possible d'être, d'atteindre l'objectif qui est proposé dans cet amendement de manière opérationnelle de créer l'indicateur sur les dossiers d'État Mining ou pas, il y a toujours de l'humain, dedans, évidemment, donc avis défavorable.

Contre. Il y a, si l'abstention, il est adopté, nous avons encore un amendement. Qui tend à insérer un article additionnel dans ce même dans cette même mission, il était également présenté par le rapporteur. Merci monsieur le président, donc le présent amendement présenté toujours par exemple François 800 au nom de la commission des finances, a pour effet de réduire le nombre des membres de la commission des infractions fiscales, le CIF de 28 à 16 conformément à la recommandation numéro 4 de la mission d'information de la commission des Finances relative à la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale, comme le relève le rapport de la mission d'information, le volume d'activité de la CIF a très fortement diminué depuis la réforme du verrou de Bercy, dans le cas de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale entre 2017 et 2021 lampe de saisine de la commission a baissé de 70 % passant de 964 saisines en 2017 à 286 en 2021 tandis que le nombre de séance et dans le même temps passé d'environ 70 à 25 d'où cette demande de baisse de des membres de la commission. Oui, merci Monsieur le Président, c'est un amendement qui fait suite à une proposition du rapport de la commission des finances sur la fraude fiscale, très bon rapport de la commission, oui c'est un très bon rapport mais il y a beaucoup de travaux sur la fraude qui sont très positifs, il y a eu évidemment les travaux de Madame Goulet et le rapport de la commission est aussi un très bon rapport et et on a, on a d'ailleurs retenu un certain nombre de propositions du rapport dans le PLF première partie et, là, dans la 2ème partie c'est un amendement qui permet effectivement de réduire le nombre de membres de la commission des infractions fiscales et je donne un avis favorable à cette proposition. Madame Goulet. on casse le thermomètre alors comme ça on est tranquille, on ne peut pas prendre la température, vu la façon et vu le nombre d'années, on a lutté pour supprimer le verrou de Bercy qu'on a seulement réussi à entrouvrir en ayant après les les les accords et les conventions pour les fraudeurs, forcément il y a moins de dossiers, moi je pense qu'il faut redéployer ses ses agents et une, et non pas supprimer les postes, quant au rapport, c'est dommage que le président Husson n'ait pas été là pour ces amendements qui tourne pas pour, pour une fois, c'est : c'est l'arroseur arrosé, parce que d'habitude, c'est les nôtres qui tourne pas alors pour une fois que c'est les siens, c'est assez réconfortant monsieur le monsieur le Ministre le le rapport de la commission des finances que j'ai lu avec beaucoup de d'attention c'est c'est ce qu'aurait dit une notre regretté doyen Weddell du plan, il parle au au à l'indicatif présent et futur, parfois au conditionnel est jamais à l'impératif, donc non moi je voterai pas cet amendement. Monsieur le Ministre. Ouvert si vous préférez l'activité de la commission s'est complètement effondré, mais les les logiquement d'ailleurs 70 % de saisines en moins, donc ça justifie qu'on fasse évoluer le nombre de membres en conséquence. Vous savez le président vénale.

je veux dire que même dans ce qui précède, il y a eu un commentaire. Pas tout à fait sûr quand même sur l'histoire, vous savez, des agents qui serait pas formés, comme nous, n'aurait pas assez pour faire les enfin de depuis quand, dans les administrations, on n'est pas capable de mobilité interne en fait tout de même allô tout ça tourne très bien. Bonsoir. Je mets donc aux voix cet amendement 438 émanant de la commission des finances, avec un avis des négatif du gouvernement favorable nous parlons favorable du gouvernement, excusez-moi et je le mets aux voix qui sont pour. D'accord, son instruction opposé. Abstention adopté et nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Crédits non répartis et nous commençons par un amendement de messieurs les rapporteurs de Montgolfier nous gêne, monsieur le rapporteur, c'est vous qui le présenter. Oui, monsieur le président, c'est c'est un amendement présenté par le co-rapporteur est Albéric de Montgolfier et moi-même, souhaitons minoré 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, le montant des crédits du programme dépenses accidentelles et imprévisible de la mission Crédits non répartis le PLF pour 2023 prévoit l'ouverture de 1 virgule 8 milliards d'euros sur ce programme, ce qui est largement supérieure au montant habituellement consacrée à cette dotation la justification invoquée par le gouvernement, qui se fonde sur les incertitudes liées à la crise énergétique et au contexte international et macroéconomique nous semble lacunaires le montant demandé nous semble en outre particulièrement excessif au regard de l'exécution des crédits de ce programme sur les exercices précédents en effet sur les exercices 2021 et 2022, aucun crédit n'a été exécuté sur cette dotation alors même qu'elle avait à chaque fois, fait l'objet à l'initiative du gouvernement et contre l'avis de la commission des finances d'une ouverture exceptionnelle de crédit en loi de finances rectificative cet amendement, s'inscrit dans une logique de sincérisation budgétaire en cohérence avec la position constante de la commission des finances sur ce sujet, la dotation conserverait, par ailleurs, un total de 774 millions d'euros, ce qui est nettement plus que les autres années en crédits de paiement, ce qui nous semble largement suffisant pour couvrir d'éventuels aléas. Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. Je crois qu'on est tous conscient qu'on fait face à un certain nombre d'aléas qui sont majeurs, on a vu ces 2 dernières années l'aléas sanitaires évidemment avec la crise Covid on a maintenant depuis près d'un an, l'aléa géopolitique avec la guerre en Ukraine, on a vu cet été, un certain nombre d'aléas climatiques. Avec des catastrophes naturelles. Donc je pense que on voit que face à tous ces risques au moment quand même de crises qu'on connaît, le fait de pouvoir disposer de fonds activable mobilisables dans l'urgence en cas de crise pour répondre à une situation d'urgence,

et d'ailleurs on a vu par le passé vous disait qu'il y avait une faible consommation, j'ai envie de dire tant mieux qu'on crame pas, entre guillemets, ces fonds là n'importe comment, mais je pense que c'est un moyen de sécurité et j'ajouterais par ailleurs que, on a renforcé les obligations d'information au Parlement, c'est la nouvelle Lolfe quand on utilise ou si on est amené à utiliser à utiliser ces fonds si on décide on décidait d'utiliser au-dessus de 100 millions d'euros de cette enveloppe, on a l'obligation de d'informer le président de la commission des finances, je le vois hocher la tête et donc c'est aussi une enveloppe qui est contrôlée plus contrôlés que les autres par le Parlement, paradoxalement, puisque quand on dépense 100 millions d'euros sur des crédits classiques ou des missions classiques, on n'a pas informé les le président de la commission des finances à chaque fois, sinon ils seraient noyés sous le travail, mais voilà donc vraiment moi je donne un avis défavorable à cet amendement parce que je pense qu'on a besoin en ce moment de sécurité. Donc Madame Goulet sweats indirectement. Faut dire que je soutiens absolument la position du gouvernement, c'est le genre de fond dont on a rêvé en matière agricole de prévention des accidents, et cetera, donc moi évidemment je soutiendrai le la position du gouvernement. Monsieur le rapporteur.

alors quand accepte 700 millions donc les les crises climatiques, il y en a déjà eu il y a la crise sanitaire, ce n'est pas rien donc ne pense pas pourquoi un milliard 8, pourquoi pas de milliards huit et l'an prochain 3 milliards ou 4 milliards non, il faut savoir s'arrêter. je précise par ailleurs que c'est des crédits qu'on n'a pas le droit de reporter d'une année sur l'autre, donc c'est quand même assez encadré et que, à chaque fois qu'on se rend compte au cours de l'année que on les on ne consomme pas une partie des crédits et qu'on en a la possibilité, on les annule on a annulé d'ailleurs dans le PLFR là le dernier PLFR on a annulé 500 millions d'euros de crédit parce qu'il restait un milliard et qu'on s'est dit bon bah on n'aura pas besoin d'un milliard dans les quelques mois qui nous séparent de la fin de l'année, donc dans le dernier PLFR on a annulé 500 millions d'euros de crédits voilà donc je pense qu'on a une gestion pragmatique de ces fonds, mais encore une fois, vu ce qui se passe en ce moment au niveau international et dans notre pays, malheureusement aussi, je pense qu'on a besoin de cette sécurité pour être réactif sous le contrôle du Parlement Oui, simplement, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je, je, je, je veux juste faire une observation à ce stade du débat et sans le prolonger mais la sincérité du du du budget et la place du Parlement, dans son exécution pour contrôler la mobilisation des crédits, même si, sur cette ligne, il y a l'autorisation des 100 millions que vous avez rappelé de façon à ce qu'on puisse avoir de vrais l'affaire avec une sincérité et des engagements de crédit qui soient, piloté par le Parlement me semble donc appeler au vote de cet amendement, merci. je mets aux voix l'amendement qui est proposée par les rapporteurs de la commission des finances, avec un avis défavorable du gouvernement, quels sont ceux qui sont pour.

donc je rappelle que je mets aux voilà amendement cette présenté par le rapporteur de la commission des finances, avec un avis défavorable du gouvernement, quelles sont les sénatrices et sénateurs qui votent pour.

adopté. Madame le Sahara. Oui. Oui merci le président cet amendement de Chantal de scène a pour but de mettre fin à une situation d'injustice dans la fonction publique hospitalière pour quelques professionnels travaillant au sein des établissements publics, sociaux et médico-sociaux principalement le secteur de l'accompagnement des personnes en situation d'handicap et de la protection de l'enfance, cause nationale reconnue si les protocoles Ségur de la santé, la fort à de la conférence des métiers ont permis une revalorisation de 189 euros Net à un ensemble de professionnels par un élargissement du complément de traitement indiciaire, une partie des agents titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière ne sont pas encore aucun argument de grade de métier de responsabilité ne justifie qu'à leurs homologues exerçant dans les mêmes fonctions à l'hôpital et on n'est pas d'bénéficient déjà de cette revalorisation depuis 2 ans, cette situation crée une différence inédite et illégitime de traitement entre professionnels relevant du même statut souvent à quelques km de distance sur les territoires, cela fragilise en conséquence les oeufs SMS concernés et la qualité de leurs services rendus, ces établissements sont peu nombreux mais cette non-valorisation salariale peut concerner jusqu'à un tiers de leur effectif aujourd'hui 3 à 4000 agents ne bénéficient pas de ce gain de pouvoir d'achat, soit 0 3 pour 100 du total des personnels de la fonction publique hospitalière, pour un montant estimé à 15 millions d'euros, le présent amendement propose un élargissement des bénéficiaires du complément de traitement indiciaire et par conséquent d'octroyer du complément de traitement indiciaire les agents administratifs, techniques, logistiques, titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière afin de respecter les existences les exigences de l'article 40, cet amendement bande de 15 millions d'euros, les exigences de l'Arctique 40, l'auteur de cet amendement était contraint de compenser la dépense par un gage sur notre programme de la mission concernés cet amendement annule par conséquent 15 millions de d'euros de l'action, du programme dépenses accidentelles et imprévisible de la mission Crédits non répartis pour les redéployer vers l'action, hein, du programme provisions relatives aux rémunérations publiques de la même mission. je demande le retrait de cet amendement, la provision relative aux rémunérations publiques regroupe des crédits ayant uniquement vocation à être répartis au sein des différentes missions du budget de l'État, cette provision ne peut donc en aucun cas être utilisé pour abonder les Budgets des hôpitaux dont le financement ne relève pas de la loi de finances de la loi de finance de la Sécurité sociale pour ça pour question de forme : demande de retrait. Je le retire, monsieur le président. Merci. Nous avons un amendement de monsieur bonhomme est signataire. Oui, c'est je vais faire vite pour monsieur PELE va le code général la fonction publique prévoit donc que les fonctionnaires résidant dans une commune où la vie est particulièrement cher, dispose d'une prime de résidence d'après les circulaires de 2001, cette prime est égale à 1 % en zone de 3 pour 100 zone hein de traitement brut de la fonction publique ah commune de résidence cette circulaire fixe également la liste des communes ouvrant droit à cette prime, or cette liste classe en général en zone de des communes où le prix de mètres carré super 25 % à la moyenne nationale soit supérieure à 3593 euros elles honneur les communes, le prix du mètre carré est supérieur à 4300 euros mais néanmoins, cette liste n'est pas mise à jour de manière automatique et aucun critère ne permet n'est clairement posé pour déterminer les communes ouvrant droit à cette prime, de fait, certaines communes, répondre à des critères formels ne sont pas inclus cette liste, c'est notamment le cas, vous avez compris pour notre collègue, elle va pour les communes de Haute-Savoie dans aucune commune les lister la circulaire, il rappelle également ce que la situation est parti humain, injuste, inégalitaire pour les fonctionnaires ou pour lesquels la situation est aggravée, donc c'est pour ça que les parlementaires de la Haute-Savoie demande depuis plusieurs années ne règle qui cette circulaire et puis ce qu'ils aillent pour le gros point de défi de de recrutement, notamment des taux de vacance de postes, notamment dans les hôpitaux, bien supérieur à moyenne nationale l'inclusion des des communes de Haute-Savoie où le mètre carré supérieur à 3593 euros représenterait un coût maximal de 5 millions d'euros ainsi cet amendement propose un transfert de 5 millions d'euros de l'action 0 1 dépenses accidentelles imprévisible du programme dépenses accidentelles imprévisible vers l'action 01 provisions dans le but d'inciter, de donner les moyens financiers gouvernement pour réviser cette circulaire. Oui, c'est un véritable problème, c'est vrai, les les logements donc de tous ceux qui travaillent dans des régions comme les stations balnéaires ou législation sports d'hiver où les logements sont très difficiles à trouver, cependant je demande le retrait de cet amendement parce que la la provision relative aux rémunérations publiques n'a pas vocation à financer cette mesure, la prime de résidence que vous évoquez, devrait notamment bénéficier aux fonctionnaires territoriaux de la fonction publique hospitalière, or les crédits du programme 551 n'vocation qu'abonder le budget de l'État, j'étais également rappeler que la provision relative aux rémunérations publiques constitue une dérogation au principe de spécialité budgétaire selon lequel écrit doit être répartis avec précision au sein des différentes missions du budget de l'État, par principe pas favorable à un recours abusif de ce à ce programme pour financer les pensions de titres de donc demande de retrait chers collègues. Très rapidement, je soutiens vraiment cet amendement parce que l'indemnité de résidence et compris perçu également par des fonctionnaires de les enseignants d'autres types de fonctionnaires, et pas seulement les fonctionnaires territoriaux et moi dans mon département, chez des communes qui qui sont parmi les communes qui ont les loyers les, les, les, les plus chers qui n'ont pas droit à l'indemnité de résiste ou les fonctionnaires n'ont pas droit à l'indemnité de résidence, alors que dans d'autres communes où finalement les, les, les loyers sont moins chers, les fonctionnaires y ont droit, donc je suis favorable à cet amendement. Donc je mets aux voix cet amendement avec un double avis défavorable, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Abstention pas adopté, nous devons voter les crédits de la mission Crédits non répartis pas de demandes d'explications de vote, la commission des finances, est favorable à l'adoption de ces crédits, je mets aux voix les crédits de la mission, ils sont ceux qui sont pour. Contre. Ils sont adoptés, il nous reste un amendement l'amendement. Sur les régimes sociaux et de retraite durant l'étape B, commençons par amendement de Madame Poncet Monge, que présente Monsieur Salmon. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, il s'agit de relever le montant de la pension minimale pour une carrière complète au niveau du salaire minimum de croissance mensuelle, c'est un amendement d'appel par lequel nous proposons donc au sein de la mission régimes sociaux et de retraite, la création d'un nouveau programme retraite minimale au niveau du SMIC pour une carrière complète, donc voilà, c'est un vrai sujet. monsieur le président, donc, cet amendement d'appel vise à ouvrir un débat sur le montant de la pension minimum sur la forme, convenons-en, cet amendement aurait plus sa place dans le cadre d'une réforme des retraites que sur une loi de finances et en tout état de cause, ce n'est pas la région la la mission régimes sociaux et de retraite qui est adapté puisqu'elle ne concerne que un nombre limité de de régime et et pas l'ensemble sur le fond, cette proposition créerait inévitablement des effets de seuil avec des pensions majorées mécaniquement au niveau du SMIC lors de la liquidation des droits sans pour autant que les pensions atteignant déjà le SMIG ou se plaçant un peu au-dessus, ne soient revalorisés de la même manière, et ainsi la valeur travail serait de fait pour partie remise en cause, c'est donc une demande de retrait. Merci Monsieur Salmon. Entendu, nous devons maintenant voter sur les crédits de la mission régimes sociaux et de retraite, la demande d'explication de vote, la commission des finances, est favorable à l'adoption de ces crédits, je les mets aux voix qui est pour. Contre. L'abstention et sont adoptés, nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial pension figurant à l'état des il y a pas eu de demande d'explications de vote, la commission des finances, est favorable à l'adoption de ces crédits, je les mets aux voix qui est pour. Qui est contre l'abstention. Ces crédits sont le encore voter sur les articles 50 et 51 qui sont rattachés pour leur examen crédit con spéciale Pensions articles 50 qui est pour. Contre adopté et article 51 même vote. Nous en avons terminé avec cette mission, l'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission Économie avec en plus l'article 43 et du compte spécial Prêts et avances particuliers organismes privés. Et pour commencer, la parole est à monsieur Thierry Cozic, rapporteur spécial de la commission des finances. Monsieur

Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, par rapport à 2022 les crédits initialement demandés pour la mission Économie augmente de 3,3 % en autorisations d'engagement, tandis que les crédits de paiement en baisse de 3,2 %. Mais la mission connaît en réalité d'importantes évolutions de périmètre pour 2023, d'une part le programme 367 financement du compte d'affectation spéciale Participations financières de l'État n'est pas abonder cette année alors qu'il était de 748 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2022. D'autre part, la mission connaît plusieurs transferts de crédits rattaché auparavant à d'autres missions pour un seul de cumuler entrant d'environ 335 millions d'euros. Au final, à périmètre constant, hors programme 367 les autorisations d'engagement augmente d'environ 520 millions, soit une hausse de 20 % et d'environ 280 millions d'euros en crédits de paiement, soit une hausse de 8,5 %. Comme l'année dernière, l'essentiel des crédits se trouve concentrée sur les moyens des grandes administrations économiques de la mission et sur 3 dispositif. Tout d'abord les compensations au groupe La Poste, au titre de ses différentes missions de service public, ensuite la compensation carbone des sites électro-intensifs dont le coût augmente d'ailleurs de 512 millions par rapport à 2022 enfin, le plan France très haut débit. S'agissant des administrations et des opérateurs de la mission tout d'abord. Leurs emplois, leur emploi et moyens sont préservés pour 2023, comme l'année dernière à appelé après plusieurs années de baisse. Concernant la DGCCRF nous sommes satisfaits de constater qu'après avoir réduit d'un quart en 15 ans ses effectifs augmentent légèrement cette année. Comme nous l'indiquions dans notre rapport, présenté il y a un peu plus d'un mois sur le sujet devant la commission des finances une légère hausse des effectifs étaient indispensables au bon accomplissement des missions de cette administration, sur l'ensemble du territoire en 2023, le plafond d'emplois augmenté de 13 opé Et ce en dépit du transfert de 60 ETPT vers la direction générale de la, de l'alimentation, c'est une bonne nouvelle, il nous faudra toutefois rester vigilant quant à l'effectivité l'effectivité de cette hausse, en cours d'exécution et aux évolutions les années suivantes. Les effectifs de la DG Trésor augmente également légèrement pour la première fois depuis 2015 hors présidence française de l'Union européenne, le plafond d'emplois augmentent ainsi 18 au BTP, tandis que son réseau à l'étranger et préserver pour la 2ème année consécutive sur ce sujet, nous avions constaté avec Frédérique Espagnac dans notre rapport du printemps 2021 que les fortes baisses d'effectifs ne pouvait continuer sans mettre en danger la diplomatie économique. Nous sommes rassurés de constater qu'elles ont pris fin. Par ailleurs, la mission est marqué cette année par l'intégration d'un nouvel opérateur désormais rattaché exclusivement au ministère de l'Économie et des Finances, il s'agit d'atout France, l'opérateur de l'État, en charge du développement touristique de la France. Il en résulte un transfert entrant de crédits dédiés à la dotation versée à cet opérateur pour environ 30 millions d'euros et de crédit destinés à développer le tourisme en France. En outre, en 2023, un effort financier est déployée en faveur des exportations et de l'interne, les internes Aziza Sion des entreprises via la hausse des subventions de Business France et de Bpifrance assurance export respectivement de 16 millions d'euros et de 28 millions d'euros. Les autres administrations ou opérateurs connaissent une légère hausse ou une stabilisation de leurs moyens, à l'exception de 2 opérateurs qui voient leurs moyens, être contraint d'une part les recettes propres de l'Institut national de la propriété intellectuelle reste plafonné à 94 millions d'euros, comme en 2022, soit un niveau qui apparaît faible, d'autre part, la Banque de France voit sa dotation se réduire de 17 millions. Frédérique Espagnac développera les enjeux liés aux politiques mises en Oeuvres dans le cas de la mission Économie dans quelques minutes je voudrais, pour ma part évoqué ici l'amendement du gouvernement intégrée au texte transmis par l'Assemblée nationale qui a rehaussé de 4 milliards d'euros, les crédits du programme 134 développement des entreprises et régulations cette hausse vise à financer une partie des 2 dispositifs d'aide aux entreprises en matière énergétique pour 2023 confirmée par le gouvernement le 27 octobre dernier pour un coût total de 7 milliards d'euros. Une hausse de 3 milliards d'euros, des crédits de la mission Écologie développement et mobilités durables vise à financer la mise en place de l'amortisseur électricité la hausse des crédits de la mission Économie de 4 milliards d'euros vise pour sa part à financer pour l'année 2023 le guichet d'aide pour le paiement des factures d'électricité et de gaz, des entreprises qui a été instaurée en 2022 de telles aides sont nécessaires et opportunes, nous resterons toutefois vigilants quant à leurs décaissements qui a été insuffisant en 2022, peut-être en raison de critères d'éligibilité trop complexe, ce sera un enjeu fort pour l'effectivité des aides annoncées. Par ailleurs, les crédits du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers, à des organismes privés s'établissent pour 2023 275 millions d'euros en autorisations d'engagement et à 495 millions d'euros en crédits de Péan je voudrais à ce propos, évoquer les prêts participatifs au profit des petites entreprises financées par le Fidesz au sein du compte du concours financier, ce dispositif a été mis en place à l'initiative du Sénat lors de la crise sanitaire, il a été prolongée plusieurs fois, ils l'offrent des possibilités de prêts aux entreprises de moins de 50 salariés qui rencontre des difficultés de financement qui n'ont pas obtenu un prêt garanti par l'État à hauteur d'un montant suffisant pour financer leur exploitation et qui justifie, enfin, de belles perspectives réelles de redressement enfin pour finir sur le sujet du compte de concours financiers nous sollicite, nous soulignons la nécessité de le dépoussiérer. En annonçant la suppression des programmes dont l'existence n'apparaît plus justifiée, en outre, la commission des finances propose donc par un amendement de supprimer le programme près avance pour le développement du commerce de l'Iran qui est un exemple parfait depuis sa création en 2018, il n'a jamais été utilisée. J'invite le gouvernement en conclusion à enclencher la suppression du programme 861 près avance pour le logement des agents de l'État dont l'utilisation est trop faible cinquante mille euros annuellement depuis 2019 pour justifier son maintien, à défaut, j'estime que ce sera au Parlement d'être à l'initiative de sa suppression, je vous remercie. Madame Espagnac vous poursuivez et vous avez 5 minutes. Je suis sûr que vous ne respecterait. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite donc en complément de mon collègue Thierry Cozic tout d'abord, aborder les compensations financée par la mission Économie versés à la Poste, outil de ces différentes missions de service public 3 compensations sont pérennisées pour 2023 tout d'abord la compensation pour financer le transport postal de la presse, par la Poste qui est maintenue et sera de 40 millions d'euros pour 2023, de même que la dotation pour le service postal universel sur l'ensemble du territoire national ne connaît pas de modifications et sera de 500 à 520 millions d'euros en 2023 enfin la dotation au fonds postal national de péréquation territoriale est maintenu pour la mission tout à fait essentiel d'aménagement et de développement du territoire de la Poste qui consiste à maintenir des points de contact dans l'ensemble du pays, en outre, en 2023 une nouvelle compensation au groupe La Poste intègre la mission Économie : en effet, la Banque Postale est chargé par la loi d'une mission d'intérêt général d'accessibilité bancaire cette mission se matérialise par l'obligation pour cet établissement d'ouvrir gratuitement à toute personne qui le demande, Livret A, fonctionnant comme un quasi-compte courant la mission vise un objectif d'insertion bancaire et social en permettant aux personnes dont les besoins spécifiques. Ne sont pas couverts par les au dispositif d'avoir accès à un support bancaires simple dont le mode de fonctionnement est adapté à leurs besoins, montant minimum de retrait faible et absence de moyens de paiement notamment cette mission représente un coût pour la banque postale qui s'explique par la consommation accrue de service au guichet en contrepartie de cette mission d'intérêt général La Banque Postale reçoit donc une compensation, celle-ci est jusqu'ici des budgétiser c'est le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations, qui en assume la charge l'article 43 du texte prévoit donc la budgétisation de cette compensation au sein du budget général de l'État, et plus précisément de la mission Économie cette réforme nous aparté nous apparaît bien évidemment opportune premièrement. Elle décharge le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations, d'une charge importante qui ne rentre pas dans le cas de sa mission principale, le financement du logement social, deuxièmement la budgétisation de la compensation, mais en cohérence l'objectif du dispositif, une mission d'intérêt général. Et le financeur, l'État pardon en outre une plus grande portée au vote des crédits par le Parlement, outre ces 2 compensation au groupe La Poste, nous avons également souhaité centre une partie de nos travaux sur le plan France très haut débit, le programme en effet 343 porte une part substantielle de la participation de l'État au financement du plan qui devrait s'élever au total à 3,64 milliards d'euros d'ici fin 2023, ce plan vise à contribuer à atteindre l'objectif d'une couverture intégrale du territoire en fibre optique à l'horizon 2025 en subventionnant les réseaux d'initiative publique les RIP qui sont mises en Oeuvres dans les zones dans lesquelles le déploiement n'est pas rentable pour les opérateurs, comme vous le savez les RIB sont des réseaux de très haut débit, mis en place dans le cadre des projets des collectivités territoriales qui doivent s'associer à l'échelle départementale pour bénéficier d'un soutien de l'État via le plan évidemment France très haut débit, il ressort de notre analyse que ce plan a eu des conséquences positives sur le déploiement du très haut débit dans les zones concernées, la dynamique est forte avec près de 1 1000000 500 1000 une nouvelle prise de fibres optiques déployées sur le 1er trimestres 2022 dans les ripe soit 64 % de déploiement sur l'ensemble du territoire dans la période, mais nous tenons évoqué plusieurs points d'alerte s'agissant du déploiement de la fibre dans les autres zones susceptibles de mettre en cause l'atteinte de l'objectif d'un déploiement de la fibre, sur l'ensemble du territoire en 2025 tout d'abord dans les zones très denses où le déploiement relève d'une initiative des opérateurs, le rythme insuffisant ces derniers pardon ces derniers semestres perdure, en outre, il existe une forte disparité entre l'avancement du déploiement dans ces zones, par ailleurs, dans les zones appel à manifestation d'investissements dit amis dans lesquelles les opérateurs privés ont pris des engagements de déploiement vis-à-vis de l'État, ces derniers ne sont pas atteints de plus, la dynamique de déploiement des opérateurs ralenti dans ces zones, enfin nos inquiétudes portent également dans les zones appel à manifestation d'engagement local les Amel, dans lesquelles les opérateurs ont également pris des engagements de déploiement sur les modèles des un avis à ce jour, seulement un tiers des locaux à rendre des locaux pardon à rendre raccordables en zone Amel l'ont été et le respect des échéances prévues dans chacun des cas n'apparaît pas assuré, bien loin de là, nous considérons donc dans ces conditions que l'Autorité régulation de l'Arcep doit impérativement se saisir de son pouvoir de sanction afin de contraindre les opérateurs à atteindre leurs objectifs, comme nous l'avons indiqué déjà l'année dernière, l'Arcep ne doit pas attendre d'être saisi par les collectivités elles-mêmes pour agir, celles-ci ne sont pas vraiment en position de force vis-à-vis des opérateurs comme nous pourrons le court, c'était sur le territoire pour lancer une procédure de sanction de la part de l'Arcep, par ailleurs, alors que des réseaux sont aujourd'hui en phase de déploiement, il nous apparaît nécessaire d'anticiper les coûts liés à l'entretien de ces réseaux, ainsi qu'à la réalisation des raccordements complexe. Le financement de ces raccordements complexe doit permettre de sécuriser l'éligibilité de tous nos concitoyens à la fibre en l'état, nous nous interrogeons sur le caractère suffisant des financements prévus, je voudrais enfin revenir sur un sujet qui concerne le Fonds de développement économique et social, en effet, il nous semble nécessaire que les conséquences du du la prolongation de l'encadrement temporaire des aides de l'État pour 2023 résultant de la décision de la Commission européenne du 28 octobre 22 soit soit pardon s'agissant du dispositif des prêts bonifiés. En effet, la décision de la Commission européenne ouvre la porte à la prolongation en 2023 du dispositif des prêts bonifiés au bénéfice des PME et ETI touchés par les conséquences économiques de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en l'état le projet annuel de performance du programme 870 cette pardon correspond pour que, cependant, ne prévoit pas la prolongation du positif, alors que des crédits non consommés demeure, ils étaient de 158 millions d'euros, l'été 2022 sur les 500 millions d'euros de dotation initiale, nous encourageons donc le gouvernement. Prolonger l'application de ce décret bonifie en 2023 en utilisant les crédits non consommés dans en 2022, sans qu'il qu'il y ait besoin d'adopter d'amendements, je vous remercie. La rapporteure. Je dois rappeler que pour cette mission, la conférence des présidents a fixé la durée maximum de discussion à 2 heures 30 en conséquence si, à une heure 30 lèveront la séance, nous n'avons pas terminé l'examen de cette mission, la suite de l'examen se réaliserait à la fin de l'émission de cette semaine ou la semaine prochaine, nous avons plus d'une heure de temps de parole dans la discussion générale et nous avons 21 amendements à débattre plus quelques votes, donc ça recommande que chacun soit attentif à son temps de parole pour des attentes pour des interventions qui ont toutes été préparées Monsieur pour la commission des affaires économiques. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon propos sera essentiellement centré sur les crédits qui concerne le volet commerce Artisanat, et consommation la mission économique on porte ceci d'étonnant qu'elle ne contient plus aucun crédit directement consacré au commerce, c'est une tendance que nous avons observé depuis plusieurs années et sur laquelle nous avions alerté régulièrement mais qui est désormais tout à fait concrètes, les annonces faites récemment par le gouvernement, censées tirer des conclusions des Assises du commerce sont par ailleurs trop frugal pour véritablement aider le commerce notamment rurales à se redynamiser la commission des affaires économiques, vous proposera donc un amendement rétablissant le Fisac afin de permettre au territoire de disposer d'arrêt l'outil utile est demandée par tous les élus de soutien au commerce, à l'artisanat, je rappelle que nous sommes passés de 25 % à 60 % de communes en France qui n'ont plus aucun commerce de proximité, c'est une situation dramatique qui pénalise l'économie le lien social et la qualité de vie de nos concitoyens, une partie des travaux de la commission s'est ensuite porté sur la situation de la DGCCRF, comme nous le savons tous ces missions sont essentiels s'accroissent avec le temps, c'est une direction centrale fondamental pour tous les secteurs qui nous intéresse, notamment en raison de son action pour lutter contre la concurrence déloyale, or elle fait face aujourd'hui à une situation ubuesque, rien que sur le dernier quinquennat trente lois et ordonnances lui ont confié des nouvelles missions devant une telle extension de son Champ de compétences, un principe élémentaire de bonne administration voudrait que ses moyens face eux aussi l'objet d'une attention soutenue du gouvernement, hé bien il n'en est rien, bien au contraire, le gouvernement et le précédent ont drastiquement diminué ses effectifs de 15 % en 10 ans, cet effet ciseau est incompréhensible et incohérent et il aboutit à des situations alarmantes dans le rapport transpartisan récent de nos 3 collègues Fabien Gay Françoise Ferrat et Florence Béatrix compta des exemples très frappant été mentionnée en matière de contrôle des informations apportées aux consommateurs la DGCCRF ne dispose plus que de 145 inspecteurs sur tout le territoire au niveau régional, cela donne un seul dans Les Hauts de France. Huit en Bretagne, sans surprise, une telle hémorragie a conduit la DGCCRF à diminuer fortement le nombre de ces contrôles, ce qui ne se fait qu'au détriment des consommateurs et des PME, certes, pour la première fois depuis longtemps 13 ETP supplémentaires sont prévus mais je regarde l'hémorragie subie depuis 10 ans, c'est l'épaisseur du trait, Monsieur le Ministre, pouvez-vous vous engager devant nous à ce que la DGCCRF puisse recruter l'année prochaine le nombre exact d'agents dont elle a besoin, en tout état de cause, la commission a adopté un amendement augmentant l'ensemble des moyens budgétaires de la DGCCRF de 5 millions d'euros voilà, mes chers collègues, les éléments que la Commission souhaitait porter à votre connaissance, je vous remercie. Madame Loisy, également rapporteur pour avis des affaires économiques. le plan France très Haut débit est désormais dotée de presque toutes les autorisations d'engagement nécessaires à sa réalisation, les objectifs sont quasiment atteint avec 82 % de locaux raccordables THD en juin 2022 soit 30 plus de 135 millions de locaux dont 75 % sont raccordables à la fibre optique, cependant, à y regarder de plus près l'activation effective des réseaux fibré n'est pas aussi rapide que le suggèrent ces indicateurs, seulement 16 un peu plus de 16 millions des foyers sont effectivement abonnés à la fibre optique, sur les 26 millions qui seraient raccordables on estime par ailleurs que 670000 foyers ne pourront être raccordés d'ici 2025 ces raccordements étant qualifiées de complexe, le gouvernement a prévu une enveloppe de 150

par an jusqu'en 2025, nous devrons donc être vigilants à ce que cette enveloppe budgétaire pluriannuel soit suffisante dans les années à venir, c'est-à-dire au PLF 2024 ces considérations budgétaires doivent être aujourd'hui appréhender au regard de la qualité du service rendu aux usagers, en effet, pour des raisons économiques, nous observons que beaucoup d'opérateurs privilégie le déploiement aérien des réseau fibré au détriment de leur enfouissement aujourd'hui, ce sont plus de 500000 kilomètres principalement situés en zone rurale qui sont ainsi vulnérables aux crises climatiques dans un contexte que nous connaissons de dérèglements de dégradation aussi de l'entretien des lignes téléphoniques ces choix économiques de court terme se font au détriment de la résilience et de la durabilité de ces réseaux stratégiques il faut Nokia, notez que chez nos voisins, comme en Allemagne, l'enfouissement et systématique, l'enfouissement des réseaux et systématique en matière de gestion des fréquences enfin l'ANFR remplit des missions croissantes dans le cas de la prospective des Jeux olympiques et paralympiques mais aussi dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi sur le renforcement qui nous tient à coeur au Sénat sur le renforcement des usages du contrôle parental sur Internet, donc les moyens de l'ANFR sont d'ores et déjà mobilisés et le feront progressivement dans les années à venir, je souligne, toutefois, Monsieur le Ministre, que la suppression de la taxe de brouillage à côté, à compter du 1er janvier 2023 et qui a été votée en fait l'année dernière et à notre sens une une mauvaise idée en tout cas, c'était un dispositif c'était un dispositif simple rapide dissuasif et il permettait effectivement à la et faire de faire appliquer la réglementation relative aux fréquences radioélectriques dont on connaît aujourd'hui toutes tous tous tous les les difficultés qui peuvent être en ont rencontré en matière de brouillage, donc nous pensons Monsieur le Ministre, qu'il serait pertinent de rétablir en fait cette amende pour brouillage dans le contexte actuel, voilà, mes chers collègues, très rapidement, les éclairages de la commission des affaires économiques. Merci pour votre exactitude cher collègue Monsieur Montaugé, rapporteur pour avis également de la commission affaires économiques la parole. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme l'an dernier, les crédits de la mission Économie représente en valeur, bien peu comparé aux montants colossaux des dispositifs du plan de relance des pays à successifs ou de France 2030, cette mission ne porte plus les moyens de la politique industrielle, en dehors de la compensation carbone des entreprises électro- intensives qui va croissant, à près de 856 millions d'euros cette année, soit environ 40 % des crédits du programme 134 c'est un effort budgétaire très significatif, auquel il n'existe aujourd'hui pas d'alternative réelle et pourtant il y a urgence à investir dans la modernisation et la décarbonation de notre industrie, d'autant que l'enjeu concurrentiel entre l'Europe et le reste du monde est exacerbée avec la pandémie derrière nous, c'est la fin des aides du plan de relance et en dehors des aides énergétiques, c'est un budget de retour à la normale qui nous est présenté pour 2023, je crains que nous n'ayons pas tirer les lotions des années que nous venons de vivre d'abord ce PLF ne prévoit aucun dispositif généraliste de soutien à l'investissement industriel qui puisse prendre le relais de ceux mis à Oeuvres lors de la relance, on risque donc un vrai creux en matière de transition industrielle par ailleurs avec la crise énergétique qui remet directement en cause notre capacité à produire en France et en Europe, il faut faire preuve d'une vision de long terme prévoir bouclier tarifaire après bouclier tarifaire ne peut pas être une réponse durable, il faut que le gouvernement contribue à la réforme structurelle du marché européenne de l'énergie, en second lieu, une plus grande résilience dans nos chaînes d'approvisionnement et de notre tissu industriel est crucial, comme notre commission là recommandé dans son rapport, 5 plans pour reconstruire la souveraineté économique je je vous soumettrai un amendement pour financer la réalisation d'une cartographie détaillée de la prise musulmane de l'industrie française et de ses vu la vulnérabilité, préalable à toute stratégie de réindustrialisation ciblées, efficaces, troisièmement, la politique industrielle bien trop concentré au plan territorial, la création de nouveaux territoires d'industrie est nécessaire, il nous faut renforcer cet outil de politique industrielle horizontale qui couvre plus largement notre territoire que les appels d'offres ciblées du PIA ou de France 2030, mon second amendement vise donc à garantir au programme territoires d'industrie un financement budgétaire pérenne sur 4 ans, enfin il ne faut pas relâcher nos efforts d'accompagnement des entreprises industrielles, au-delà de la crise qui semble être derrière nous, je vous proposerai donc un 3ème demain pour renforcer les moyens de Business France car il me semble essentiel d'accentuer l'effort d'internationalisation des entreprises industrielles françaises en cette période charnière porteuse de risques mais aussi d'opportunités en conclusion, j'aimais au nom de la commission, un avis favorable sur la mission économie que je conditionne toutefois l'adoption des 3 amendements que je viens d'évoquer, je vous remercie. Et pour la commission de l'aménagement du territoire, le développement durable, monsieur Jean-Michel Houllegatte, rapporteur pour avis. Que le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a émis un avis favorable sur les crédits relatifs à l'aménagement numérique du territoire de la mission économique ont pris dans le programme 343 France très haut débit, cependant, le déploiement de la fibre optique constitue cette année, un sujet sur lequel la Commission lance également un appel à la vigilance, en particulier sur 3 points qui ont déjà été évoquées premièrement si l'objectif d'une couverture en fibre de 80 pour 100 du territoire fin 2022 est en bonne voie et le fort dynamisme des déploiements en zone d'initiative publique laisse espérer une atteinte de la cible, dans un futur proche, le ralentissement des déploiements zone d'initiatives privées, lui, est inquiétant, le nombre de logements rendus raccordables a par exemple chuté de 54 % par rapport à 2021 en zone d'appel à manifestation d'intérêt et de 47 % en zone très dense, je rappelle que la zone est couverte en fibre, qu'à 87 %, alors que les opérateurs devaient initialement assurer une couverture intégrale pour fin 2020 si les pouvoirs publics ne dispose pas de levier d'intervention en zone très dense, le régulateur et ça déjà été mentionné l'Arcep a la responsabilité de rappeler ces opérateurs aux engagements qu'ils ont pris s'agissant de cette zone appel à manifestation d'intérêt en ayant recours à ses pouvoirs de coercition, si nécessaire, deuxièmement sur les raccordements complexes comme il a déjà été dit 150 millions d'euros ont été prévues par le gouvernement pour apporter une rallonge financière via un mécanisme d'appels à projets aux collectivités territoriales en zone d'initiative publique ces moyens supplémentaires sont nécessaires, mais loin d'être suffisant, les raccordements complexe caractérisée par un manque de génie civil sur la partie terminale de raccordement représenterait de un à 2 millions de prises et des besoins dépassant le milliard d'euros, surtout la pertinence même de cet outil est sujette à interrogation, monsieur le Ministre, plutôt qu'un appel à projets ne serait-il pas préférable d'instituer un dispositif de financement pérenne permettant une péréquation entre les territoires, conformément aux principes fondateurs du plan France très haut débit, enfin sur la résilience des réseaux numériques une réflexion doit également s'engager sur les effets du dérèglement climatique sur les réseaux fibre qui sont majoritairement installés comme ça, elle a été déjà indiqué par voie aérienne, plus largement, il nous faut anticiper les dépenses liées à l'exploitation et à la maintenance des réseaux qui sont particulièrement élevés en zone d'initiative publique, or le plan France très haut débit ne prévoit pour l'heure, aucun mécanisme de solidarité financière entre les territoires, sur ce point, les déploiements des réseaux progressant, il s'agit à présent de réfléchir aux actions nécessaires pour assurer leur fonctionnement dans la durée que vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Nous pouvons engager la discussion générale, et la première intervenante et Madame. Daphné Ract-Madoux qui a la parole pour six minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission, Économie et à ce titre, je tiens à saluer le travail de qualité réalisés par nos collègues rapporteurs spéciaux, Thierry Cozic et Frédérique Espagnac, tout comme celui d'Anne-Catherine Loisier de Serge Babary et de Franck Montaugé, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et Jean Michel pour la commission Développement durable et Aménagement du territoire, ce travail est déterminant à l'heure où le Parlement joue plus que jamais un rôle vital cette mission permet de mettre en oeuvre des réformes décisives pour la compétitivité de notre économie, pour favoriser l'emploi et dessiner les contours d'une vision économique stratégique, elle est le rouage clé permettant le fonctionnement à plein régime de la locomotive France sur les rails de l'économie mondialisée, avec près de 3 9 milliards d'euros, cette mission, qui se veut ambitieuse, voit néanmoins ses crédits de paiement baissé de plus de 3 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2022 avec mes collègues de l'Union centriste nous saluons cependant la poursuite de l'effort de soutien à la modernisation de l'économie et à sa transformation écologique et numérique, la mise en oeuvre du plan France 2030 la montée en charge de l'Agence nationale des fréquences ou encore l'attribution de moyens conséquents pour soutenir des entreprises électro-intensives sont autant de témoignages des ambitions qui sont celles de notre pays à ce titre, mes chers collègues, je tiens à m'attarder sur 3 dispositifs qui me semble fondamentaux pour l'avenir de notre économie, premièrement la crise énergétique impliqué une réponse à la hauteur des enjeux, les 360 millions d'euros supplémentaires dédiés aux mécanismes de compensations de carbone en faveur des entreprises électro- intensives mises en oeuvre par là des jeux sont ainsi cruciaux pour pallier les effets des hausses du prix de l'électricité, nous devons nous en féliciter, face à la crise énergétique et aux inconnus qu'elle emporte nous devons accompagner nos entreprises pour leur donner des garanties et maintenir carnet de commandes et compétitivité, deuxièmement, la stabilisation des crédits et des employes de la DGCCRF est à saluer, pour continuer de bénéficier de services efficace et performant en 2023 son plafond d'emploi augmentera de 13 ETP, conformément aux recommandations de la mission de contrôle sénatoriales formulées en 2022 mais l'ajout de 5 millions d'euros supplémentaires en autorisations d'engagement grâce à un amendement de notre de nos rapporteurs est un signal fort vers la sanctuarisation des moyens de la direction. Enfin, Business France joue depuis de nombreuses années un rôle décisif pour accompagner nos entreprises sur les marchés internationaux, dans l'attente de nouveaux contrats d'objectifs et de moyens signé avec l'État, il était indispensable d'envoyer un message clair à nos entreprises, en renforçant les moyens de cet acteur clé à l'heure où notre balance commerciale est plus que jamais déséquilibré, c'est chose faite avec les crédits de cette mission et le travail de nos rapporteur de la commission des affaires économiques, avec une hausse de plus de 15 millions d'euros après 4 années de baisse à titre complémentaire, je soutiens pleinement l'amendement du rapporteur prévoyant d'ajouter 8 millions d'euros pour consolider les moyens dédiés à l'accompagnement de la transformation numérique de nos entreprises, si les ambitions de cette mission sont donc à saluer et que nous la voterons nous sommes loin de la carte blanche, ainsi attirer votre attention sur 3 points qui appelle votre vigilance sur le plan France très Haut débit : tout d'abord dans les zones peu denses, les engagements ne sont pas tenus les crédits ne sont pas au niveau pour les zones amis et Amel ça la 2 a déjà été dit, le compte n'y est tout simplement pas mes chers collègues, c'est la compétitivité des territoires qui est en jeu : l'Arcep doit se saisir de son pouvoir de sanction pour assurer le déploiement optimum des réseaux et l'atteinte des objectifs, cela passe par des moyens adaptés et un soutien infirmer cette mission à un parent pauvre, les chambres de métiers de l'artisanat, elles voient leurs ressources diminuer de près de 15 millions d'euros dans ce PLF à travers une baisse du montant de recettes de la taxe pour frais de chambre des métiers qui passerait en l'état de plus de 200 millions d'euros à 188. Ce n'est ni acceptable ni envisageable ces chambres joue un rôle décisif dans la promotion de notre artisanat d'excellence, véritable vitrine de la santé économique de nos territoires, nous avons d'ailleurs voté ce matin à la quasi-unanimité, un amendement permettant le maintien de leur crédit et je forme le voeu qu'ils soient conservés dans le texte final, j'en profite pour dire tout mon soutien à l'ensemble des réseaux consulaires dont il faut sanctuariser les ressources car il joue un rôle décisif et accompagne quotidiennement et en proximité le développement de nos entreprises, enfin, en dehors des crédits exceptionnels liés aux enjeux énergétiques, les crédits ordinaires liés à l'industrie au sein de la mission se situeront en 2023 à un niveau similaire ou inférieur à celui des années précédentes, je suis certaine que le ministre-Lescure en cette semaine de l'industrie partagera le fait que ce n'est pas une bonne nouvelle à l'heure où nos organisations syndicales et patronales, tire la sonnette d'alarme quant au risque de plus en plus grand de désindustrialisation de notre pays, vous l'avez compris avec mes collègues de l'Union centriste nous saluons la vision stratégique qui est la vôtre, tout comme les crédits attribués pour faire face aux défis énergétiques à la réforme de la poste ou pour promouvoir nos entreprises à l'international, cependant, nous devons continuer, ambitieux tant en matière industrielle que numérique, à l'heure où ces défis structurels conditionneront la compétitivité de notre pays et de son économie, c'est donc avec vigilance et exigence que nous voterons cette mission je vous remercie. Madame panthères la parole pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame, monsieur, les rapporteurs, mes chers collègues, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2023 nos échanges, nos échanges pardon s'inscrivent dans un contexte atypique, les impacts de la guerre en Ukraine et les conséquences de la crise sanitaire ont un retentissement certain sur les données conjoncturelles au niveau régional, national, européen et international, nous avons toutes et tous conscience dans cet hémicycle, et nous le mesurons au contact des artisans, commerçants et chefs d'entreprise de nos territoires respectifs, l'augmentation des prix de l'énergie, les problèmes d'approvisionnement qui handicape la production et les intentions d'investissement sont revus à la baisse par crainte d'une aggravation de la situation, l'évolution des crédits de la mission Économie suit inévitablement à ces phénomènes, ce qui doit au préalable être saluer l'effort financier d'un Suchard, oh combien important doit répondre aux besoins du tissu économique et notamment au secteur du secteur de l'industrie pourvoyeur d'emplois de qualité et contribuant au dynamiques locales au sujet du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, nous reconnaissons les bienfaits qu'il a pu apporter ces derniers mois et ces dernières années aux structures touchés par les crises nous observons comme les rapporteurs une forte variation, variabilité du solde d'une année à l'autre, mais cela s'explique en grande partie par le fonctionnement pluri-du compte, il met en exergue des prix dans le remboursement est lissée sur plusieurs années, nous comprenons donc il s'agit, hein, partie de dispositifs répondant à des besoins identifiés sur une période de borné dans les 7 programmes concernés ne partageons l'avis des rapporteurs spéciaux sur le numéro 861 en effet, les 50000 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sans quelque peu anecdotique et montre une pertinence relatif de continuer à les faire figurer dans cette section ça naturellement, remettre en cause l'utilité d'un tel, outil d'accompagnement au sujet du programme 862 il nous paraît particulièrement significatif tard il constitue un véritable filet de sécurité, il permet en effet à l'État d'octroyer des prêts ponctuels aux entreprises ah Restructuration et rencontrant des difficultés à accéder au marché du crédit via le Fonds pour le développement économique et social nous soutenons donc le maintien des 75 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement aussi nous avons approuvé l'amendement des rapporteurs qui vise à prolonger donna le dispositif des prêts participatifs pour les petites entreprises de portage également la volonté de suppression du programme 868 sur le développement du commerce avec l'Iran qui était totalement anachronique, notamment en cette période où l'on constate une forte répression du régime des mollahs iraniens sur la population et en particulier sur les femmes, par ailleurs, une discussion a eu lieu sur le programme 869 des prix à la société concessionnaire de la liaison Express entre Paris et l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle, les 200 millions d'euros en autorisations d'engagement pour couvrir les surcoûts du nouveau report de la livraison des travaux et les 348 4 millions d'euros en crédits de paiement pour suivre le rythme de décaissement de près interroges au-delà de l'intérêt du projet que nous ne remettons nullement en cause l'explosion des coûts et le non-respect des délais de mise en service de l'infrastructure sont clairement à déplorer, nous resterons donc vigilants quant à son avenir, pour que cela ne continue pas éternellement grever le budget d'année en année enfin, au sujet des autres programmes comme les prêts octroyés dans le cadre des Investissements d'avenir, nous n'avons pas d'observation supplémentaires au regard du fait qu'ils suivent des trajectoires ordinaire, en somme, le groupe du Rassemblement démocratique et social européen porte un regard favorable à cette version du compte de concours financiers, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole maintenant Madame Micheline Jacques pour les républicains, avec 5 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je vous prie d'excuser Monsieur Patrick Chaize, qui aurait dû intervenir en discussion générale et qui m'a demandé de le remplacer la mission Économie est aujourd'hui un ensemble de crédit disparates et dispersées, qui n'est plus représentatif des politiques économiques menées aujourd'hui désormais largement financé par des crédits et des mesures extra-budgétaires, ce qui nuit d'autant plus à la clarté des débats au contrôle parlementaire du budget de l'État parmi cet ensemble de crédit sans grande cohérence, je note toutefois de points d'intérêt le 1er concerne la compensation des déficits des 4 missions de service public du groupe La Poste, pour 2021, le coût Net cumulé de ces 4 missions est évaluée à 1,69 milliards d'euros pour un niveau cumulé de compensation de 1,12 milliards d'euros dans 250 millions d'euros pour le service universel postal 174 millions d'euros pour la contribution à l'aménagement du territoire, 88 millions d'euros pour le transport et la distribution de la presse et 338000 millions d'euros pour l'accessibilité bancaire, les montants sont élevés, mais ils sont à la hauteur de l'importance des services publics postaux comme le rappelait le rapport d'information, de Patrick Chaize Pierre lourd et Rémi Cardon, si nous nous satisfaisons des compensations budgétaires pluriannuels pour ces 4 missions de service public, les incertitudes demeurent pour les années à venir sur la mission de contribution à l'aménagement du territoire, la baisse des impôts, de production et la suppression progressive de la CVAE doivent être prises en compte, c'est le cas dans le PLF 2023 une compensation budgétaire complémentaire d'environ 66 millions d'euros sera nécessaire dans la paix dans le PLF 2024 afin de maintenir le niveau de la compensation, je rappelle qu'il est vital de pérenniser les 17000 points de contact postaux sur le service universel postal, les modalités d'attribution du bonus de 20 millions d'euros doivent être clarifiés rapidement au regard de l'entrée en vigueur de la nouvelle gamme de services pour ce poste au 1er janvier 2023 dans le PLF pour l'année 2021, le gouvernement a fait le choix d'accorder par défaut, ce bonus, alors même que les indicateurs de qualité de service n'était pas connu la qualité de service n'est pas une option, c'est une exigence, une demande des collectivités territoriales, des entreprises et des usagers dans les manques mécontentements sont réels, il y a un autre domaine dans lequel la qualité de service est primordial, c'est celui des télécommunications, ce qui m'amène au 2ème, point d'intérêt de cette mission Économie les avancées du plan France très Haut débit 100 satisfaisante et les objectifs devrait globalement être atteint d'ici 2025 la France demeure tout de même le 1er pays de l'Union européenne en matière de déploiement des réseaux fibré, même si certaines parties de notre territoire 113 en marge de ces déploiements en particulier Mayotte à cet égard, nous disposons de très peu d'informations sur les moyens financiers alloués au nouvel appel à projets visant à développer les réseaux d'initiative publique dans ce département, encore trop éloignées des politiques publiques dans certaines zones et sur certains réseaux ancien, la qualité de service n'est pas au rendez-vous, les mécontentements sont réels et le secteur des télécommunications, manque d'un régulateur fort et exigeant, sommes-nous en train de confondre vitesse et précipitation, le plan France très Haut débit est dotée de toutes les autorisations d'engagement nécessaires à sa réalisation, nous devons donc désormais faire très attention à la qualité du service rendu, c'est l'objet de 2 propositions de loi que Patrick Chaize a récemment déposé la première relatives à la qualité à la pérennité des réseaux et la seconde, relative à l'entretien des lignes téléphoniques d'un point de vue budgétaire, l'enjeu se situe désormais au niveau du financement des raccordements complexe leur bonne réalisation permettra à la fois l'atteinte des objectifs du plan France très haut débit et la bonne fermeture du réseau cuivre à l'horizon 2030, si une enveloppe de 150 millions d'euros est prévu sur 2 ans, les besoins sont plutôt estimé à 300 millions d'euros par an jusqu'en 2025, je reçois joint ainsi notre rapporteur Anne-Catherine Loisier car nous devrons veiller à la reconduction d'une enveloppe budgétaire suffisante au financement des raccordements complexe au delà de 2023 en jeu il y a l'accès au très haut débit jusqu'au dernier mètre et jusqu'au dernier abonnés je vous remercie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente, mes chers collègues, la mission économique que nous examinons aujourd'hui détermine une partie des moyens que l'État consacre au développement économique de notre pays, ils sont notamment destinés à favoriser l'emploi, la croissance, la compétitivité des entreprises et le développement des exportations, on peut constater que les crédits de cette mission, pour 2023 sont en hausse, elle porte 3 ambitions : la première consiste à un soutien à l'économie et à ses acteurs pour faire face au contexte international et national, réside réside dans la poursuite de l'accompagnement vers la transformation numérique écologique de notre économie et le 3ème est caractérisée par l'ajustement de nouveaux dispositifs de régulation adaptée aux réalités, l'examen de cette mission m'amène à faire quelques remarques, je peux tout d'abord déploré la disparition du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce Fisac c'est regrettable car c'est un instrument d'une grande utilité pour nos territoires, il est le principal outil d'accompagnement des évolutions des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services, il permet de financer des opérations portés par les collectivités territoriales ou les chambres consulaires ainsi que les actions individuelles d'entreprise artisanale dans les dans les, dans je soutiens donc pleinement l'amendement déposé par le rapporteur Serge Babary, dans le cadre du programme 134 est adopté par la commission des affaires économiques, qui prévoit l'oncle le déblocage de 30 millions d'euros pour établir ce dispositif qui concourent largement à la préservation et au développement du tissu d'entreprises de proximité concernant le sort réservé aux chambres des métiers de l'artisanat, ce texte entendait amputé donc des ressources des CMA à hauteur de 15 millions d'euros pour atteindre un objectif de 60 millions d'euros en 5 ans. Nous pouvons que donc cette véritablement un mauvais signal pour se pour un réseau consulaire qui ont accompagné, donc les entreprises pendant la crise, les aide à affronter au quotidien les difficultés et les épaules en terme de succession et de reprise. Toujours plus sollicitées pour la mise en place, donc de différents programmes tels que Action coeur de ville, les CMA subissent ainsi les conséquences de la hausse du coût de l'énergie à laquelle on peut aussi ajouter donc celle de la masse salariale du fait de la revalorisation du point d'indice concernant donc les avancées portées par cette mission, je voudrais souligner la forte hausse des crédits consacrés à la compensation carbone des sites et des entreprises électro-intensives, elle s'élève à 856 millions d'euros, cette augmentation devrait se poursuivre dans les années à venir, ces entreprises sont bien évidemment très consommatrice d'énergie et sont particulièrement exposés d'urgence dans cette crise énergétique inflationniste, la France compte plus de 500 entreprises et qui emploie 90000 personnes dans un secteur ô combien stratégique cette compensation est absolument indispensable pour la compétitivité de la filière, maillon essentiel de notre souveraineté industrielle enfin après des années de baisse, les moyens de la DGCCRF sont en progression, je voudrais donc le saluer et l'amendement adopté en commission, qui tend à augmenter les moyens de la DGCCRF de 5 millions d'euros ce notamment cela vient corriger donc l'absence de corrélation entre l'augmentation de ses missions et de son Champ de compétences et la baisse de ses moyens, en effet, depuis une dizaine d'années, elle, elle doit faire face donc à une baisse de ses effectifs évalués à environ 15 en conclusion et au regard des avancées introduites le groupe les indépendants votera en faveur de l'adoption de cette mission ainsi qu'amender et permettez-moi donc en mot de conclusion également de saluer le travail de nos rapporteurs. Merci, cher collègue, la parole est à Monsieur Daniel Salmon.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, mes chers collègues, le budget consacré cette année à la mission Économie très représentatif d'une politique court- termisme du gouvernement composé de mesures disparates conjoncturelle et curative, une politique qui continue à aider en priorité les grands gros les grandes promesses d'après-Covid d'aller vers une plus grande résilience de notre système productif et de notre tissu économique et industriel ne sont pas là, le gouvernement a retenu dans le texte sur lequel elle a engagé sa responsabilité un amendement augmentant de 4 milliards d'euros, les crédits du programme 134, ceci afin de financer la compétitivité des entreprises électro-intensifs, face à la hausse du coût de l'énergie, montant qui n'est pas sans poser question par son poids au sein de la mission, comparé à d'autres secteurs d'activité également impacté par la crise, avant de revenir sur ce sujet, permettez-moi d'abord d'analyser ici les crédits initialement demandés pour 2023 à périmètre constant, hors programme 367 les autorisations d'engagement augmente de 20 % et les crédits de paiement de 8 5 % une hausse, mais une hausse en trompe l'oeil liée en grande partie à l'augmentation de la compensation carbone pour les entreprises et à la rebudgétisation des prestations réalisées pour l'État par la Banque Postale auparavant, financé par la Caisse des dépôts, quant au commerce et à l'Artisanat, comme le soulignait notre rapporteur pour avis, ils sont les parents pauvres de cette mission, plus aucun crédit ne venant abonder ces secteurs phares pour l'économie de nos territoires, c'est pour cela que nous proposerons un amendement visant à rétablir le Fisac qui jouait un rôle central pour lutter contre la désertification économique et commercial en zone rurale et contre la dévitalisation du centre-ville, il a apporté des aides ponctuelles et ciblées dans un objectif de complémentarité, voire de rééquilibrage des une action locales parfois insuffisantes faute de crédits disponibles, nous posons également un point d'alerte sur la DGCCRF alors que ses missions de plus en plus complexes se sont démultipliés, ces dernières années, le gouvernement refusait de lui octroyer les moyens humains et financiers pour assurer ses objectifs d'intérêt général, pire encore, elle a vu ses effectifs fondre en perdant près de 1000 agents en 15 ans si les 13 TP prévus dans le PLF sont bienvenues et permettent de stopper l'hémorragie, ils sont clairement insuffisants, nous soutiendrons vivement les amendements visant à lui octroyer des crédits supplémentaires qui sont un 1er pas afin d'amorcer enfin nous l'espérons, une nouvelle dynamique pour cette administration, notamment pour la protection des consommateurs, j'en reviens aux crédits relatifs à la industrie une part massive de crédits alloués à la mission économique va donc servir à la compensation carbone des sites électro-intensifs au total 856 millions d'euros financeront 500 sites pratiquement 150 pour 100 de plus par rapport à la et les montant auquel il faut ajouter les 4 milliards du nouveau dispositif de soutien, si l'on entend bien entendu la nécessité d'assurer le maintien des capacités de production, on peut néanmoins s'interroger sur le niveau de cette hausse exponentielle qui s'accroît d'année en année et l'accumulation de dispositifs d'aide pour des entreprises qui ont un impact écologique très important pourtant il faudrait là aussi amorcé une réelle transition et orienter l'action publique plutôt dans l'accompagnement de la transformation de nos modes de production, de consommation et vers la sobriété énergétique en ce sens, le budget de l'État doit soutenir davantage, entre autres, l'économie sociale et solidaire, un modèle de référence pour l'économie de demain à travers le respect des écosystèmes et le partage de la valeur au service du bien commun, un soutien bien plus massif doit être entrepris pour en faire un outil de résilience de l'économie dans les territoires, en conclusion, si nous seulement la préservation globale des crédits, la mission Économie ne perds mettras ni de créer des emplois, ni de faire progresser nos entreprises dans la voie de la bifurcation écologique, hélas, nous n'avons toujours pas pris la mesure de la gravité de la situation.

Bien Monsieur le le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, madame madame mesdames et messieurs les les rapporteurs souveraineté économique, c'est un terme qui était au coeur de nos débats, il y a quelques semaines, c'est un terme d'ailleurs que le président de la République, dès 2017 dans ce moment, discours de la Sorbonne avait employé depuis lors il y a eu véritablement cette volonté de reprendre le contrôle sur un certain nombre de politiques économiques, industriels et cette mission porte une partie, une partie seulement parce que, naturellement, d'autres crédits sont dans France relance dans France 2030 en tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est un accroissement significatif de ces crédits c'était mentionné à l'instant même plus 1 % alors même s'il y a l'augmentation importante de la compensation carbone poser trop intensif mais ça participe de cette politique industrielle et donc on peut s'en s'en féliciter, je crois que ce qu'on peut voir dans dans l'évolution des crédits de de cette mission, et singulièrement je m'attarde un peu plus sur le problème 134 c'est le fait que le gouvernement, l'État a toujours été là en soutien dans les crises, de façon très conjoncturelle, mais également de façon plus structurelle dans une forme de réarmement si je puis dire, soutien dans l'urgence parce que les plans de résilience, on avait été porté par cette mission, et puis on l'a vu l'amendement massif de 4 milliards d'euros, qui était adopté pour mettre en place justement les différentes aides le guichet d'aide pour faire face au choc des prix de l'électricité, et puis il y a également ce qui a l'internationalisation Business France qui reçoit 15 millions d'euros supplémentaires, ça va permettre de développer un certain nombre de programmes, les vitrines de faire venir des acheteurs internationaux en France, ça fonctionne très bien et puis naturellement, hé bien contribuer à ce que les sujets liés aux services au tourisme notamment, puis trouver à à continuer sur leur lancée avec le plan de reconquête dont les crédits sont sanctuarisés, en partie dans cette, dans cette mission et j'aurai un mot peut-être pour l'événementiel, on y reviendra à l'occasion d'un amendement, mais qui doit également continuer à être accompagné de façon plus générale au-delà de ce soutien ponctuel, dire que le réarmement, il passe par le fait que, il y a un coup d'arrêt à la fin de la baisse des effectifs d'un certain nombre de services, c'est vrai dans la DGE, par exemple, plus 19 ETP et ça signifie aussi d'ailleurs que nous devons nous appuyer sur les réseaux consulaires et et c'est pourquoi ce matin, effectivement, nous avons été un certain nombre à à voter l'amendement en faveur des chambres de métiers de l'artisanat puisque comme les CCI sont des vrais relais sur le terrain du fait de la disparition de près de 275 emplois ces dernières années dans le réseau des concentrés de la DGE et puis la mission elle porte également tout ce qui a trait la transformation école écologique et et numérique, le plan France très haut débit, regardons, vous venez d'où on vient, en 2020 19 millions de locaux raccordés en FTTH, on en est à 32 millions il faut voir le chemin parcouru, voilà, le diable est dans les détails, il faut aller jusqu'au dernier kilomètre au dernier maître ah dernière porte mais je crois que c'est un très beau succès d'ailleurs, la France est le pays dans lequel, en Europe on déploie le plus de fibres, très clairement, voilà, ça, ça participe de cet aménagement du territoire, au même titre que la Poste et comme d'autres orateurs je je me félicite que le Front national du péréquation territoriale soit toujours là soit toujours abondé, et puis peut-être un petit mot pour pour dire que, effectivement, il faut ne pas délaisser ni la consommation ni le commerce et, de ce point de vue là je salue la création effectivement d'effectifs à la DGCCRF, là aussi, venant mettre un coup d'arrêt à une baisse depuis 15 ans hein, donc on voit bien tout ça n'est pas d'hier, et dire que du coup les crédits supplémentaires ah DGCCRF doivent faire en sorte que on ampute pas les crédits dédiés aux associations locales de consommateurs, ça a été une tentation par le passé et donc je veux absolument prévenir de ce point de vue là et puis sur le commerce, c'est vrai, le Fisac, il avait un vrai rôle pour l'instant, il y a pas encore encore tout à fait la la version de substitution, il est très important, là aussi, d'aider les commerces à faire face à la digitalisation pour qu'il puisse lutter à armes égales, on a aussi des sujet d'équité mais également qui puisse faire face aux enjeux de sobriété énergétique, on sait qu'il y a le décret tertiaire qui est devant nous, hé bien, pour tout ça il y a besoin aussi d'être armé et donc d'ailleurs des politiques et monsieur le Président, je terminerai, on voit bien les limites de la main invisible du marché, donc moi je salue, hé bien la main visible de l'État qui est là pour structurer accompagner les filières économiques de notre pays grâce aux crédits de la mission que le groupe des pays votera. Merci, cher collègue,

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après les interventions des rapporteurs j'aimerais au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain vous donner notre appréciation globale sur l'ensemble du projet de budget de la mission économique dans la loi de finances pour 2023, nous étudions ces crédits de la mission, Économie, dans un contexte de retour inédit de l'inflation, notre collègue Franck Montaugé bien d'exposer dans ce contexte, l'utilité de la compensation carbone des entreprises électro-intensives, c'est un effort massif mais néanmoins indispensable cependant notre rôle de parlementaires et de voir et d'anticiper, au-delà de la conjoncture immédiate, l'enjeu majeur pour notre économie, particulièrement pour notre industrie et l'investissement technologique et matériel dans la décarbonation, la compétitivité de demain est conditionné à la sortie du terme fossiles quels outils budgétaires et public, mettons en place au service du renouveau des politiques industrielles et pour l'accélération des transitions énergétique comment prolonger l'effort nécessaire initiée par les crédits du plan de relance avec des outils, des moyens adaptés, y compris pour les PME et pour les ETI, cela n'a, paraît pas clairement à la lecture du budget on ne je ne vois pas aussi fortement. La main visible de l'état que mon collègue, si nous voulons que notre économie recouvre sa souveraineté industrielle sa position industrielle, nous ne devons pas manqué de relever ces nouveaux défis, nous devons tirer les leçons d'hier qui ont conduit à désindustrialiser désindustrialisation que nous payons très cher, très cher en témoignent d'autres déficit du commerce extérieur abyssal, cette année, ce déficit catastrophique dépassera 150 milliards d'euros, donc il s'agit pour nous de retrouver des spécialisations industrielle compétitive décarbonnées c'est une première étape essentielle, donc, outre les politiques macro-économiques visant à accroître la compétitivité, la question de l'efficience des, des dispositifs de soutien à l'exportation se pose notre collègue Franck Montaugé évoqué à juste titre, à la nécessité de renforcer les moyens de Business France le précédent contrat d'objectifs et de moyens entre cette agence et l'État a conduit à une baisse de financement de Business France au cours de ces 5 dernières années, cela a été composée, nous dit-on, par divers financements exceptionnels dans le cadre des mesures d'urgence, puis via du le plan de relance, il n'en demeure pas moins que le financement global de Business France n'est pas à la hauteur, surtout si on se compare aux pays étrangers, en particulier à nos homologues européens, le rapport de la Cour des comptes sur Business France de 2021 est à cet égard édifiant le différentiel de financement public et quasiment de A4 entre Business France et son homologue britannique, l'agence italienne bénéficient quant à elle, le double de financement public que Business France la Cour des comptes relève également nonce un récent rapport d'octobre 2022 sur les dispositifs de soutien à l'exportation que le contrat d'objectifs avec l'État incite Business France à maximiser ses recettes, principalement via les cette recherche de ressources pénalisent la mine la mise en oeuvre. D'une stratégie basée sur des priorités sectorielles et géographiques, elle pénalise aussi l'accompagnement des entreprises dans la durée, un financement public plus large à la hauteur de nos homologues européens, et donc indispensable afin de rendre cette politique de soutien plus performante en matière de chiffre d'affaires réalisé à l'export. Autre domaine qui nous tient à coeur les crédits liés à la consommation, ils ont attiré toute notre attention dans la droite ligne du rapport que nous avons réalisé avec mes collègues Fabien Guez Françoise Férat, en juin dernier sur l'information consommateurs je souhaite donner écho aux propos du rapporteur Serge Babary concernant la DGCCRF, alors que les et que ses effectifs ont baissé de 15 ans depuis près de 10 ans, nous soutenons l'amendement de la commission visant à augmenter ses moyens. Concernant maintenant le l'Institut national de la consommation et les associations de consommateurs les moyens des uns des autres sont depuis des années, très malmené, ils contribuent pourtant largement et régulièrement alerter les consommateurs sur les risques et dangers, ils sont dans leur diversité, un facteur important de formation d'information de nos concitoyens, il y a urgence à les soutenir davantage, enfin, vous me permettrez d'achever mon propos en évoquant la situation générale de l'économie sociale et solidaire, je dois regretter que la feuille de route ministérielle sur l'ESS à la suite du séminaire gouvernement-gouvernementale de cet été ne soit pas suivi d'effets budgétaires suffisantes dans le projet de loi de finances 2023 dans le cadre des travaux de notre groupe d'étude ESS au Sénat, nous avons pu constater le manque de moyens des crèches pour développer l'ESS dans nos territoires, nous proposerons un amendement afin d'y remédier, j'ajoute, en août, que nous avons besoin pour l'avenir d'un document budgétaire en mesure de retracer l'effort de l'État en faveur de toute l'économie sociale et solidaire, ça permettrait un pilotage plus fin, plus sûr et nous avons déposé avec mon groupe, plusieurs amendements pour se soutenir ce activité ce activité économique très important qui fait montre d'une grande résilience, j'ajoute que le ESS est vraiment un acteur de transformation, un pan de une filière de transformation écologique, économique, sociale de notre pays, c'est un formidable creuset d'innovation sociale, soutenons la plus fortement, je vous remercie. Merci, cher collègue, monsieur Fabien Gay. La parole pour le groupe communiste, écologiste et citoyen.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos nombreux rapports autour de scandales sanitaires Lactalis les graines de sésame, les faux steaks et bien d'autres, ou encore notre rapport sur l'information aux consommateurs ont tous clairement pointé dans notre diversité politique, le manque de moyens de la DGCCRF, surtout que la multiplication des missions confiées sans moyens supplémentaires viennent aggraver cette situation pourtant la décision de renforcer son Champ d'intervention au numérique et de la doter d'un pouvoir de sanction plus étendue, ont constitué des avancées très importantes qui ont permis d'amplifier son action de régulateur de l'ordre public économique, je le dis parce que c'est une nécessité, Dave inventer ses capacités aux nouveaux défis de l'économie ah ces mutations et en particulier celles issues de l'ère digital et numérique, qui se développe à grande vitesse, c'est une décision nécessaire et bienvenu envoie hanches et vous le voyez venir il y a un mais qui n'est pas négligeable lorsqu'on regarde le projet de loi de finances que vous proposez, c'est le recul des moyens de la DGCCRF et je parle de recul en toute conscience, malgré les 13 emplois temps plein qui sont ajoutés à ses effectifs parce que lorsqu'on ajoute des missions qui sont complexes chronophage, il faut être clair : soit on ajoute des moyens suffisants pour qu'effectivement un nouveau Champ de compétences soit développées effectif, soit on ne lui donne pas les moyens nécessaires pour assurer à la fois ses missions traditionnelles et ces nouvelles prérogatives et cela signifie qu'on reste sur un effet d'annonce qui ne se concrétisera jamais et là je suis désolé de le dire, mais 13 emplois temps plein supplémentaires, ce n'est même pas ce dont la DGCCRF a besoin pour ses missions habituelles, je ne vous donne pas ici une interprétation personnelle, je vous parle, avec des chiffres qui sont sans appel et je vomissais remercie d'ailleurs nos collègues, rapporteur de la mission Économie pour leur exposer clair et limpide, la DGCCRF a perdu 15 % de ses effectifs en 10 ans, 15 pour % alors que dans le même temps, le commerce en ligne se développe à vitesse grand V 100, alors que de nouvelles formes d'activité économique difficile à réguler vient de créer de nouvelles formes de pratique commerciale trompeuse qu'il faut absolument combattre aujourd'hui la DGCCRF n'a pas les moyens pour assurer ses missions, vous avez un espace hors des lois hors du temps parfois avec les contenus éphémères sur les réseaux qui permet de l'activité économique illégale sans conséquence pour ses auteurs, et là je vous parle du numérique, mais le manque de moyens, la DGCCRF, c'est un drame pour tous les secteurs de notre économie, pour celles et ceux dont les TPE-PME respectent les règles mais subissent une concurrence déloyale aussi nos agriculteurs comme les vignerons français avec l'usurpation d'appellation pour nos associations aussi, rappelez-vous aussi du scandale des faux sec, il y a 3 ans, mais surtout pour les consommateurs et consommatrices qui doivent s'y retrouver dans une surenchère permanente de la Belle de publicité ou d'emballage trompeur imaginer que, dans le Lot, c'est un seul agent qui travaillent sur ces questions, mais aussi pour la sécurité, la conformité des produits comme l'ont démontré les nombreux scandales alimentaires avec la multiplication des accords de libre-échange assurément là des DGCCRF aura du pain sur la planche pour vérifier la conformité des produits alimentaires, aujourd'hui nous sommes précisément au moment où les mots doivent devenir des faits, c'est l'attente que doit satisfaire ce projet de loi de finances et en l'état les ambitions qui sont affichés sont loin d'être concrétisé et je note que pour la première fois, le rapporteur a proposé une hausse de 5 millions que je soutiendrai mais je proposerai, chers collègues, si vous en êtes d'accord de rajouter 20 millions supplémentaires pour que cette mission s'exerce dans l'intérêt général, je vous remercie.

ma première remarque concernant la mission Économie aura trait à sa forme, elle agglomère des crédits particulièrement disparates qui tantôt finance le fonctionnement de certaines directions comme l'Insee, la DG Trésor ou la DGCCRF, tantôt des actions comme la compensation carbone l'achat d'études économiques, la gouvernance des pôles de compétitivité, le service public postal et etc, on observe à la lecture de cette mission de fortes hésitations quant à la politique économique à mener bien entendu je n'ignore pas que d'autres missions du budget général concourent également à la mise en oeuvre des politiques économiques, mais il me semble qu'en matière de présentation du budget, la clarté est primordiale pour nos concitoyens et ce n'est pas le cas tout d'abord, il y a une forme de trompe l'oeil dans cette mission, en apparence, et si l'on se fonde sur la version initiale, les crédits de la mission augmente de 860 millions d'euros, ce qui est une bonne chose, mais en réalité, un tiers de la hausse provient de la simple rebudgétisation des prestations réalisées pour l'État par la banque sociale et près la Banque Postale, pardon, et près de 50 % de la hausse sont liés à l'augmentation de la compensation carbone, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de réels efforts en matière de soutien à l'économie, de fait, cette mission est surtout devenue le support des actions du gouvernement pour soutenir les entreprises face à la hausse des coûts de l'électricité, c'est la raison pour laquelle le gouvernement il y a ajouté 4 milliards d'euros de crédits à l'Assemblée n'a Sonia national pour financer les entreprises les plus consommatrices d'énergie en matière énergétique, le constat établi par la commission des affaires économiques n'est guère engageant les montants alloués au volume d'énergie sont insuffisants et aucun dispositif structurel n'est avancée, les dernières mesures annoncées laisseront encore trop de petites entreprises dans la détresse, la situation des industries électro-est hyper électro-intensives n'est pas meilleure aujourd'hui nos concurrents hors UE dispose une visibilité à 25 ou 30 ans, et peuvent se fournir en électricité à Bakou, autant qu'il le souhaite, permettez-moi d'insister sur la situation de l'industrie française car elle est particulièrement préoccupante, nous payons le prix fort, d'une perte de souveraineté économique qui résulte de mauvais choix politiques et de l'inaction du gouvernement depuis plusieurs années, les annonces des récents plans de relance, plan de résilience et France 2030 ne concerne qu'un nombre trop faible d'action et n'engage pas de mesures suffisamment structurante pour l'avenir, en 2023 les crédits ordinaires liés à l'industrie au sein de la mission Économie se situeront à un niveau similaire voire inférieur à celui des années passées, aucune aide directe pour le secteur industriel n'est prévue, à l'exception de financement résiduel des pôles de compétitivité et de la compensation carbone, cette dernière est la principale aides directes portées par la mission depuis plusieurs années, mais elle ne sera pas soutenable, il apparaît urgent d'investir massivement dans la technologie de décarbonation de l'industrie pour rééquilibrer la concurrence entre l'Union européenne et les pays étrangers, s'agissant des aides à l'innovation et à l'investissement, elles sont portées par les programmes d'investissements d'avenir successifs et par le plan France 2030, je le regrette, dans la mesure où cet éclatement des moyens ne permet pas de définir une fois de plus, une politique industrielle claire à long terme par ailleurs et comme l'a souligné, notre rapporteur les PIA et France 2030 sont déployés à travers des appels d'offres nationaux difficilement accessible pour nos PME et nos ETI, cela est d'autant plus regrettable que la conjoncture économique demeure incertaine et que les transformations industrielles s'accélère, il manque une vision de long terme pour que la France puisse regagner en compétitivité rééquilibrer sa balance commerciale et défendre sa souveraineté industrielle protéger nos industries en adoptant des mesures structurantes, c'est faire le choix de l'indépendance de la France en conservant la maîtrise de nos matières premières dans des secteurs indispensables pour la transition énergétique, par ailleurs, je me réjouis de l'adoption par la commission des affaires économiques, d'un amendement permettant d'augmenter les moyens budgétaires de la DGCCRF, en effet, comme nous l'expliquer tout à l'heure notre collègue rapporteur Serge Babary : comment faire plus avec toujours moins avec des moyens qui ne le permettent pas, enfin les travaux du rapporteur pour avis sur le financement des associations de consommateurs me semble important, et il sera intéressant de connaître vos intentions en la matière, monsieur le Ministre, force est de constater que le nombre d'associations nationales agréées, conduit à un saupoudrage des subventions publiques et la diminution des subventions entamé il y a quelques années, se fait selon des critères pour le moins obscures ainsi je formule le voeu que le gouvernement puisse nous éclairer sur l'ensemble de ces sujets et je vous remercie.

il m'appartient de rappeler les priorités qui sont les nôtres, tout en m'efforçant de répondre aux principales observations que vous avez formulées dans cette discussion générale qu'procéderait en 3 temps : le 1er étant consacré aux mesures de soutien à l'économie, le deuxième à sa régulation et le troisième aux comptes spéciaux de prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés dans la conjoncture difficile que nous connaissons le soutien aux acteurs économiques reste notre priorité pour l'année 2023, comme l'ont rappelé les rapporteurs spéciaux, Thierry Cozic et Frédérique Espagnac ce soutien prend principalement 3 formes d'abord les aides aux entreprises en matière énergétique sont amplifiés, nous poursuivons notre politique d'accompagnement des entreprises électro-intensives au travers du dispositif de compensation carbone dans un contexte où la compétition internationale s'intensifie, je pense notamment à l'inflation oui d'Auxonne Act américain, qui est une véritable menace pour l'industrie française et européenne, cette considération liées à la compétitivité de nos entreprises se doublent, bien sûr, d'un souci environnemental de plus avec la forte tension sur le prix des énergies les guichets d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité ouvert à l'été 2022 sont reconduits simplifié et élargi en 2023 et je vous rejoins monsieur le rapporteur sur le fait que les critères était évidemment trop restrictif, nous étions en cela aussi encadré encadré au niveau européen, mais nous allons avancer notamment avec l'amortisseur électricité dédié aux PME et TPE qui complète le dispositif qui couvre ainsi l'ensemble des acteurs économiques, le soutien que nous apportons à l'économie passe aussi par un effort accru pour permettre l'accessibilité universelle aux services postaux bancaires et numérique ça été rappelé notamment par Frédérique Espagnac ce soutien vise tout d'abord des missions essentielles, assuré par la Poste, c'est dans cette perspective qu'ont été intégré au budget général de l'État pour 2023, le financement de la mission d'accessibilité bancaire à hauteur de 303 millions d'euros le financement du service universel postal pour 520 millions d'euros, ainsi que la hausse de la subvention à la mission d'aménagement et de développement du territoire, l'accès au réseau de fibre optique répond également à cet enjeu d'aménagement en permettant à nos concitoyens, aux entreprises et aux collectivités qui s'y raccordent de bénéficier de la qualité de service du très haut débit je suis sensible aux attentes légitimes d'une démarche encore plus volontariste en termes de déploiement, je voudrais rappeler que le programme France très Haut débit répond avant tout à des besoins connu les crédits inscrits pour 2023 en montant de 437,7 millions d'euros sont donc adaptés aux perspectives de déploiement sur le terrain et inclut un appel à projets spécifiques pour Mayotte, je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir dans les amendements, en parallèle, nous poursuivons notre objectif d'amélioration de la compétitivité des entreprises par des soutiens ciblés la souveraineté industrielle et numérique n'est pas un slogan, c'est un objectif qui requiert un effort constant pour assurer la compétitivité de nos entreprises, les dispositifs French Tech destiné à favoriser la croissance en France et à l'international des Start-Up ou d'escalope et France num dédiée à l'accompagnement de la transformation numérique des PME, TPE complète efficacement l'appui apporté aux régions dans la gouvernance des pôles de compétitivité pour le maintien et le renforcement de l'investissement et l'innovation dans les filières industrielles et technologiques, enfin, nous continuerons d'accompagner les entreprises exportatrices à travers le soutien offert par Business France dont le budget a été renforcée de 15 millions d'euros et BPIFrance l'intégration d'atout France dans la mission Économie réaffirme s'il en était besoin l'importance des secteurs du tourisme et des petits commerces dans la vitalité de l'économie française, ces derniers sont également soutenus par les dispositifs Action coeur de ville et Petites Villes de demain et par des dispositifs du plan de relance son fonds de restructuration des locaux d'activité manufacture de proximité sur le Fisac, monsieur babary, vous l'avez abordé, j'ai eu l'occasion, indiqué dans les débats du PLF qu'un dispositif équivalent qu'une enveloppe dont l'objectif se rapproche de ce qui était le Fisac figurera dans le fond vert que nous allons mettre en place et qui figure au PLF d'une façon générale, les orientations évoquées décrivent clairement nos priorités protéger largement des chocs externes offrir un socle commun de services sans discrimination territoriale et soutenir des démarches plutôt que des catégories d'acteurs, la 2ème, chose que je veux souligner c'est que l'émission de régulation de l'économie sont renforcés dans ce projet de loi de finances, au regard de l'effort de soutien à l'économie que nous engageons en 2023, les outils de prospective de régulation, de contrôle et de suivi doivent être performant, c'est pourquoi les emplois et les moyens des administrations et opérateurs de la mission Économie sont préserver, voire renforcer ses ressources vont permettre à l'Insee de poursuite de la modernisation de ces outils statistiques à l'Agence nationale des fréquences, la capacité de piloter le déploiement de la 5 G et des réseaux de fibre optique d'accompagner les nouveaux usagers et d'accroître l'information des des citoyens sur cette technologie nouvelle à l'autorité de la concurrence de poursuivre son développement et je veux répondre à Madame Loisier sur l'ANFR et sur la taxe brouillage effectivement c'était une taxe qui était utilisé comme sanction, ce qui n'est pas tout à fait l'objectif d'une taxe, c'est la raison pour laquelle elle s'arrête, mais la direction générale des entreprises, je vous l'annonce : travail, un mécanisme de sanctions qui pourra prendre le relais et je demanderai que vous soyez tenus informés de ses travaux, bien évidemment, je souhaite évoquer à présent le cas de la DGCCRF, dont les missions sont essentielles pour la protection des consommateurs, et pour la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale pour 2023 la DGCCRF bénéficient donc de 84 créations d'emplois, j'ai entendu monsieur Guey, parler de 13 créations d'emplois, 13 c'est le plafond d'emplois, le plafond d'emplois et relevé de 13 ETP, mais il y a ensuite le schéma d'emplois c'est différent et le schéma d'emplois c'est quatre-vingts IV, créations d'emplois à la DGCCRF 50 pour assurer les contrôles relatifs à l'accessibilité des biens et services pour les personnes en situation de handicap et 34 TP afin de couvrir les besoins d'accompagnement de la livraison et l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 en parallèle la DGCCRF voit son Champ d'intervention rationaliser, avec le transfert de la mission de sécurité alimentaire qui donne lieu à la création de 90 emplois à la direction générale de l'alimentation, en plus des 60 emplois transférés ce ne sont pas 60 agents qui quitte la DGCCRF au 1er janvier 2023 mais le transfert de missions se déroulera en parfaite Intelligence entre les de direction la DGCCRF continuons évidemment d'assurer l'accompagnement de la DGAL dans cette nouvelle mission, enfin le dernier point que je veux mettre en exergue, c'est que le compte spécial de prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés et ramener un fonctionnement classique avec la fin de la crise sanitaire, en effet, l'accompagnement des entreprises en difficulté au cours de la crise Covid 19 avait requis l'ouverture d'un dispositif public d'octroi d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés auxquels ont été ajoutés les prêts exceptionnels aux petites entreprises et le fonds de transition, l'ensemble est clos en 2023 mais je précise que les entreprises auparavant éligibles pourront se voir proposer des prêts à taux bonifiés ne demeure donc actif en 2023 qu'un prêt à la société concessionnaire de la liaison Express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, le fonds pour le développement économique et social qui attribue les financements de l'État à des entreprises pour accompagner leurs restructuration financière et commerciale, et enfin le dispositif avance aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement s'il n'est doté que de 50000 euros, ce dispositif demeure pertinent manifestement et garantit un État réactif en facilitant et en accélérant la prise de fonction des agents servant à l'étranger pour la par l'attribution d'une aide voilà Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, ce que je pouvais vous dire rapidement parce que nous n'avons un temps limité, en réponse à vos interventions, mais nous allons maintenant échanger sur les amendements, merci. portant sur les crédits de la mission Économie figure aller taper, nous commençons par un amendement 191 qui sera présenté par Madame Pentel, je suppose. 191. Monsieur le président merci l'activité de l'ensemble des entreprises de l'événementiel professionnel, organisateur sites d'accueil et prestataires de service. Au salon congrès réunion d'entreprise a été particulièrement impactés depuis mars 2020 les fermetures et restrictions administratives pendant quasiment 18 mois ont provoqué une perte de chiffre d'affaires, les besoins d'investissement de la filière sont pourtant toujours plus fort, d'une part les défis environnementaux pèse sur des investissements de la filière, les sites événementiels sont appelés à mettre en oeuvre ou leur transition énergétique, il leur rénovation thermique dans le cas de la modernisation de leur espace d'accueil, or l'épuisement de leurs fonds propres, là les empêche de faire face à ses ambitieux programme d'investissement, d'autre part, les événements internationaux que notre pays s'apprête à accueillir d'ici à 2024 nécessite une mobilisation de l'ensemble de la filière leur bande leur bonne organisation risque d'être compromise par la vulnérabilité de la trésorerie des acteurs de la filière, ainsi que la hausse des coûts de l'énergie, cet amendement vise donc à accorder à ces entreprises du secteur événementiel professionnels dans les critères d'éligibilité seront définies par décret, des instruments de quasi-fonds propres, à un taux proche de l'OAT, avec une liberté d'usage merci. Merci, cher collègue, alors nous sommes obligés de faire la présentation des 13 amendements en série, c'est la loi de la la loi procédurale de discussion commune et donc nous serons reconnaissants le rapporteur, de bien vouloir donner sa vie dans l'ordre pour qu'on puisse ensuite voter à peu près éclairés donc ensuite Madame Berthet, qui présente l'amendement 43. merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la sécurisation du plan d'alimentation des entreprises en énergie est cruciale pour la continuité de leur activité économique, leur compétitivité et le maintien des emplois dans de nombreux secteurs, seuls les gaz peuvent apporter les puissances en pointe nécessaires à l'activité économique et de nombreuses entreprises souhaitent d'ores et déjà sécurisé sur le moyen terme leur approvisionnement, une baisse de 7, approvisionnement en gaz naturel peut donc faire craindre quant à la pérennité de ces entreprises et des emplois associés, il est néanmoins possible d'investir dans des équipements de secours de substitution temporaire alimentés au propane et à terme au bio propane néanmoins la crainte de ne pas utiliser ses équipements et de réaliser un investissement inutile empêchent souvent les entreprises de franchir le pas, ainsi, je vous propose par cet amendement que ces investissements puissent être déduits de liesse l'année de leur réalisation, il permettrait de soulager les réseaux électriques et gaziers pour passer les pics de consommation, d'assurer la continuité énergétique sur l'ensemble du territoire en limitant la prise de risque d'investissement de stabiliser les émissions de de CO2 en offrant une solution alternative à la substitution du gaz naturel Vert le fioul, d'autant plus que les équipements installés pour le propane sont compatibles avec le bio propane, il s'agit de permettre aux entreprises de se fournir en énergie cet hiver et de préparer l'avenir, ces mesures sont cohérentes avec le plan de sobriété, présenté par le gouvernement, cependant, les règles de recevabilité m'oblige à gager via un transfert de crédits provenant à regret d'une autre, d'un autre programme de la mission. le précédent, les seules choses qui les différencie sur des impacts budgétaires merci. Ensuite, monsieur Montaugé, au nom de la commission d'amendement 89. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre et cher, cher collègue. Près près de 4 ans après sa création, on constate que le programme territoires d'industrie et est devenu un instrument efficace de politique industrielle horizontal et qu'il est apprécié TAM par les élus locaux, que les chefs d'entreprise est considéré comme un un cadre important de de dialogue et de soutien au au pro aux projets territoriaux donc dans le cadre du du plan de relance, je, je rappelle que ce programme a au déploiement des volets territoriaux des dispositifs nationaux du type plan de relance, près d'un milliard d'euros d'aide de l'État et les régions ont pu être ainsi mobilisés pour aider et accompagner 1800 projets industriels au coeur des territoires français bon cependant les les financements spécifiques qui ont été dégagées dans le contexte de la relance, arrive à échéance à la fin de l'année 2022, et voilà le le gouvernement a annoncé la prolongation du dispositif mais sans forcément le le doter de de nouveaux financements spécifiques et pourtant le le besoin et là sur les territoires, il y a des projets, il y a des élus qui veulent accompagner les porteurs de projets industriels, donc il faut il abondé une ligne spécifique de financement du du programme territoires d'industrie, donc on le propose à travers une enveloppe budgétaire de 5 millions d'euros sur 4 ans la là une ligne, une ligne spécifique dans le dans le programme 134 une ligne qui pourrait s'appeler donc territoires d'industrie tout simplement qu'il n'existe pas, à ce jour, je précise que cet amendement a été voté à l'unanimité en en commission des affaires économiques. Merci, ensuite le 207 présenté par Madame, l'actrice compta. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, donc dans mon intervention tout à l'heure j'ai indiqué que Business France manquèrent réellement de moyens, notamment si on le compare assez. Nos homologues européens et Business France a besoin de davantage de financement public pour développer ses moyens d'action sa mission de soutien à l'internationalisation. Des entreprises françaises, notamment industriels, on se rend compte par exemple que certaines entreprises n'exporte qu'une fois et c'est quand même regrettable que ces entreprises ne soit pas à nouveau, donc il y a vraiment un soutien à mon avis, il y a un amendement de la commission a eu 8 millions d'euros en soutien de Business France mais personnellement je pense qu'il faut aller nettement de la pour se rapprocher des financements publics octroyés par nos homologues européens, leurs agences de soutien à l'exportation que Business France soit moins contraint de rechercher des ressources propres et travaille à une stratégie en termes géographiques en termes d'entreprises ciblées pour l'exportation, donc c'est le sens de cet amendement, c'est vraiment de donner à Business France les moyens pour mieux accompagner nos entreprises à l'export parce que on a un déficit, cela a été rappelé, on aura un déficit du commerce extérieur très important cette année, il y a une part conjoncturelle il y a une part liée à la compétitivité, mais il y a aussi une part liée à l'accompagnement des entreprises, je vous remercie. Merci ensuite monsieur Babary pour l'amendement 87. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, cet amendement vise à réinstaurer le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce fameux Fisac et le doté de 30 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au sein de l'action 23 du programme 134 Développement des entreprises et régulations outils de soutien de secteurs du commerce et de l'artisanat mal, notamment dans les zones rurales le Fisac important progressivement été mis en gestion extincteurs puis totalement supprimé à compter de 2021 or, de l'avis général des différents acteurs élus locaux fédérations de commerçants réseau consulaire et cetera cette suppression est regrettable à plusieurs titres, d'autant que la dévitalisation commercial de nombre de territoires s'aggrave et pénalise les collectivités leurs habitants comme l'a montré un rapport sénatorial conjoint de la commission des affaires économiques et de celle de l'aménagement du territoire et du développement durable, publié en mars 2022, en effet, 59 % des communes françaises ne dis dispose plus d'aucun commerce de proximité, alors qu'elles n'étaient que 25 % en 1980 bien qu'imparfait, ce levier, confie une certaine latitude aux élus locaux pour sélectionner les projets commerciaux, artisanaux qui souhaitaient voir mis en oeuvre dans leur territoire et tu as entendu qui sont les plus aptes à avoir une vision globale et partagée de son aménagement, en outre, si des dispositifs de soutien au commerce existe sur d'autres formes, il présente plusieurs inconvénients : le programme Petites Villes de demain reste récent le programme Action coeur de ville ne concerne que les villes moyennes, les régions n'ont pas une connaissance fine de dynamique commerciale et artisanale, il est proposé par conséquent d'abonder l'action vingt-trois d'une somme de 30 millions d'euros. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre collègue Serge Babary a déjà donné de nombreux éléments puisque cette mon amendement est le même : je compléterai juste avec quelques quelques éléments également la mise en extinction du Fisac donc en 2019 reste en travers de la gorge, de nombreux maires, pourquoi donc arrêté à un outil qui donnait la possibilité, pour les communes d'être les financeurs Directs des commerçants, c'est en contradiction totale avec la politique nationale en faveur de la revalorisation des centre-et des centres bourgs, les programmes Action coeur de ville ou Petites Villes de demain ne concernent finalement que peu de communes et ne répondent pas spécifiquement aux besoins d'aide du commerce et de l'artisanat, dans les territoires ruraux c'est pourquoi cet amendement comme le précédent, vise à restaurer le Fisac qui a le doté de 30 millions d'euros, j'ai bien entendu le Ministre tout à l'heure, mais je dirais à un tiens vaut mieux que 2 tu l'auras, dans le fond Vert merci.

problèmes de nouvelles techniques de communication et qui a pour objet, cet amendement, le financement du projet très haut débit à Mayotte amendements élaborés aussi en concertation avec notre collègue Thani Mohamed l'objectif final du plan France très haut débit, le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de bout-en-bout sur l'intégralité du territoire, le département d'outre-mer, avait en effet des problématiques spécifiques à gérer problématique que ne connaissent pas les autres départements en métropole, de ce fait, ce après avoir rattrapé une partie de son retard d'aménagement numérique suite au raccordement de Lille via un 1er câble sous-marin, notamment en recours dans les principaux sites techniques par le biais d'une dorsale de collecte optique, le département de Mayotte enfin pu travailler son à son projet 100 % fibre cependant malgré les mais les conditions de ce plan s'étant considérablement restreinte depuis 2002 18 Mayotte qui aurait pu initialement bénéficié de 27 millions d'euros de ce plan, voit sa subvention théorique descendre à 4,5 millions d'euros dans la version liée au plan de relance afin que l'histoire ne se répète pas, et que Mayotte puisse pleinement s'inscrire dans ce plan, quel qu'il a été conçu à l'origine, cet amendement donc 22,5 millions d'euros d'autorisations d'engagement, ce qui permettrait une subvention à la prise de 540 euros par ligne donc ce cet amendement et aussi de surtout dans une démarche d'équité territoriale, merci.

Des baisses des effectifs depuis 10 ans, on est d'accord tous ensemble, que 400 ETP ont été perdus en disant : ça fait 6 ans que vous êtes aux affaires, la traduction. C'était qu'en 2010 il y avait aucun département qui comptait moins de 8 TP aujourd'hui 2021, les chiffres de 2021 14 départements. Au moins de 6 ETP et 38 en au moins dix ça, c'est les chiffres, alors après vous ancrer 84 très bien cinquante sur des nouvelles missions et 34 sur les Jeux olympiques, alors j'ai une question Monsieur le Ministre est-ce que ces agents seront pérennisés après 2024. Et où seront-ils réattribuer et la 2ème chose vous avez parlé des 60 agents. Qui vont partir à la DGA, le parce que c'est eux qui vont s'occuper maintenant de la sécurité alimentaire. Imaginons, monsieur le ministre. Il y aurait 20 volontaire. Il y aurait 20 volontaire et donc il y en aurait 40 qui voulait pas partir est-ce qu'ils seront considérés en sur, effectif. Et ce qui se et est-ce que. Pour le coup, cela aurait une conséquence sur les concours de recrutement en septembre 2023 je vous remercie. Il y a une mutation d'office de ensuite monsieur pour l'amendement 88. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, il s'agit également d'un amendement sur la DGCCRF telle que je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit d'un constat amplement documenté largement déploré le nombre de tâches, confiée à la DGCCRF augmente d'année en année ces moyens ne suivent pas, ce qui ne peut qu'aboutir une situation sous-optimale en matière de protection des consommateurs, le contrôle de la conformité des biens, services et de la régulation de la concurrence ainsi sur les 5 dernières années 30 loi ailleurs de Lens sont venus compléter l'émission dont la DGCCRF à la charge en parallèle les moyens techniques, financiers et humains juridique et cetera de la DGCCRF n'ont pas augmenté et ont même baissé depuis plus de 10 ans, ce qui ne peut que conduire à diminuer le nombre de contrôles ou abandonner certains pans de son activité au profit de dossiers jugés prioritaires entre 2010 et 2021 le nombre d'établissements visités est passé de 160000 à 91000, et le nombre de visites effectuées a diminué de 238000 à 134000, cette situation n'est plus tenable alors que les actions de la DGCCRF devront encore se multiplier dans les prochaines années à mesure que le la réglementation environnementale entre en vigueur et donc proposé d'abonder l'action numéro 24 d'une somme de 5 millions d'euros. Merci, cher collègue, ensuite c'est madame Jasmin qui présente son amendement 196. Merci monsieur Monsieur le Ministre, depuis le 1er février 2022, les règles de dédouanement ont changé et c'est dorénavant la Poste qui s'en charge, en lieu et place des services de douanes si ce changement n'est pas en soi un problème : les tarifs les quand même réclamé au moment de la récupération des colis suscite la colère des usagers ultramarins les sommes représente en effet entre 30 et 50 % de la valeur du produit commandé ainsi entre la TVA, l'octroi de mer régional et les frais de livraison par voie aérienne, la facture est salée et a du mal à passer auprès des usagers en colère, l'objectif de cet amendement et de mettre en place une péréquation tarifaire des colis postaux équitable, incluant les outre-mer, cela relève d'une des missions de service public dans le cadre du monopole confié à la Poste en outre-mer dès lors les segments où les coûts sont de plus faible viennent financer les secteurs ayant un coût plus élevé pour présenter un coup uniforme à l'ensemble des usagers, c'est in fine et le principe de solidarité nationale qui s'avère d'autant plus important pour les territoires d'outre-mer, notre amendement propose donc de majorer de ces millions d'euros, la dotation budgétaire versée à la Poste, soit 1 % du montant de la dotation annuelle totale qui s'élève pour 2023 à 500 millions d'euros pour assurer le service public dans des conditions plus acceptables pour les outre-mer je vous remercie. Merci madame monsieur Barnier, encore un, l'amendement le 188. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre le présent amendement a pour objet d'augmenter de 3 millions d'euros, les crédits de l'action 23 industries et services du programme 134. Développement des entreprises et régulations afin de financer le lancement d'un chèque pour la transmission d'entreprise, reprenant la proposition 9 du rapport Reprendre pour mieux entreprendre dans le territoire, présenté par messieurs Michel qui Calvez Rémi Cardon Olivier Rickman est adopté à l'unanimité par la délégation aux entreprises en octobre 2022, le rapport de la délégation, a mis en évidence l'un des obstacles à la transmission d'entreprise en France, qui est le manque d'anticipation et d'accompagnement des dirigeants de TPE et PME or désormais 25 % des chefs d'entreprise ont plus de 60 ans j'ajoute 11 % ont plus de 66 ans jusqu'à 700000 entreprises seront à transmettre dans les 10 prochaines années, c'est pourquoi, afin d'encourager les dirigeants entre 55 et 65 ans à mieux anticiper le devenir de leur entreprise, la délégation propose que leur soit proposé à chèque pour la transmission d'entreprise permettant de financer les coûts relatifs à la valorisation de l'entreprise, le conseil juridique, la réalisation d'audits financiers, sociaux ou environnementaux pour établir un diagnostic lancement en 2023 pour réviser un chèque de 3000 euros pour environ 1000 bénéficiaires surtout TPE et petites PME, je vous remercie. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, la protection à la défense des consommateurs constitue une politique mise en oeuvre par un ensemble d'acteurs, les associations, dont la présence territoriale est essentiel, bénéficie de la pluie de centres techniques régionaux de la consommation et de l'Institut national de la consommation, qui sont de véritables plateformes de proximité en leur apportant ressources alors que les informations n'ont jamais été aussi nombreuses impliquant davantage de contrôles, on l'a vu les effectifs de la DGCCRF ne sont pas suffisants et il en va de même pour les fonds alloués aux associations de protection des consommateurs, la Cour des comptes dans un rapport rendu en 2021 évoque une diminution globale des subventions aux associations agréées de 40 % alors que le rôle de vigie n'est n'est plus à démontrer, le rapport d'information que nous avons commis avec Fabien Gay Françoise Férat sur l'information du consommateur, souligne à quel point cette situation incompréhensible, n'est pas tenable et qu'il faut renforcer la protection du consommateur, donc une des recommandations était de renforcer les effectifs de la DGSE DGCCRF mais aussi de mettre fin à la baisse des dotations aux associations de protection de consommateurs et donc dans un contexte de contraction du pouvoir d'achat avec des mutations qui s'opèrent les sites, les citoyens sont parfois démunis, ils ont besoin de nouveaux repères et donc notre amendement a pour objet de de Jade interroger le gouvernement sur sa politique en matière de protection des consommateurs et quels moyens il entend allouer et enfin pour cet exercice de renforts de réaffirmer l'importance du rôle des associations et d'ajuster leurs moyens en conséquence, je vous remercie. Très bien, donc maintenant madame et monsieur le rapporteur, si vous voulez bien nous donner des avis de la commission, en commençant par le 191. Merci monsieur le président, donc sur le l'amendement 191 qui a été présentée par Madame planté l'amendement propose de d'accroître le programme 134 de 500 millions d'euros en fait en faveur du secteur élevé de Montiel et en en effet c'est un secteur qui a été fortement affaiblie pendant la crise sanitaire, en dépit des moyens publics qui ont été mobilisés à la lecture de de l'amendement, nous constatons que tout dispositif d'aide envisagée devrait néanmoins être conforme au droit européen en matière d'aides de l'État. ce que la que les rapporteurs font sur cet amendement, c'est une position de de retrait nous qu'on ne nous interprétons ce cet amendement comme un amendement d'appel pour le gouvernement. Merci monsieur le président si vous m'autorisez, je je ferais le le 43 et le 192 puisque il s'agit du du même amendement donc qui vise à la création de nouveau programme intitulé prévenir le maintien, l'activité économique, même en cas de rupture d'approvisionnement énergétique temporaire nous ne partageons l'esprit de de de cet amendement sécuriser l'alimentation des entreprises en l'énergie et notamment en gaz est essentielle, en revanche, il nous semble que financer avec l'argent public, l'achat d'équipements de secours de substitution temporaire n'est pas ce qu'il a de plus vertueux pour la dépense publique, le montage que vous proposez par ailleurs avec une aiguille diction dièse sur les dépenses engagées et davantage bon fiscal que budgétaire, donc c'est une demande de retrait pour les deux le 89 sur l'ouverture des lignes budgétaires doté son millions d'autorisations d'engagement en faveur du dispositif territoires d'industrie cet amendement adopté par la commission des affaires économiques concernant un sujet important sur la réindustrialisation de nos territoires, le dispositif territoires d'industrie créé en 2018 et porteur d'un peu moins de de 2000 projets ce sur l'ensemble de notre territoire, a été jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à présent doté de financements divers dont les fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires doté de près de 1 milliard d'euros, vous souhaitez monsieur Montaugé par votre amendement crée une ligne spécifique au sein du programme, c'est entre quatre enfin de ce dispositif de front pérenne pour un total de 100 millions d'euros en autorise monde en autorisation parlons d'engagement, nous partageons bien évidemment la nécessité de soutenir la la réindustrialisation des territoires, néanmoins, cela ne peut se faire au prix de financement du programme 305 Stratégie économique, il en a également besoin il revient finalement au gouvernement de créer des financements ou de lever le gage, Monsieur le Ministre, nous vous interrogerons donc sur le devenir du du dispositif du dispositif territoires d'industrie je précise-t-il personnel, je suis favorable Monsieur Montaugé à votre amendement, donc nous sommes mais ben non, avis de sagesse, pardon, excusez-moi. Alors, ensuite, nous sommes là, l'amendement 207. L'amendement 207 présenté par Madame Blétry compta, donc c'est un c'est une proposition de d'une hausse de 50. Millions d'euros des crédits dédiés à Business France le soutien aux exportations et à l'Internet 2 internalisation des entreprises françaises et notamment porté par la mission Économie il y a de subventions celle à Business France et c'est la BPI France assurance exporte la subvention à Business France sera en 2023 de 100 millions d'euros, en hausse de 15,6 millions d'euros, soit environ 18 % néanmoins cette hausse doit être relativisée, elle fait suite à plusieurs années de baisse. Depuis 2020 Business France bénéficient de crédits conséquents provenant du plan de relance, ce qui ne sera plus le cas en 2023, une partie des 15,6 millions d'euros supplémentaires prévus en 2023 sera mis en réserve dans ce contexte, augmenter la subvention apparaît pertinent, mais le montant proposé par cet amendement, à savoir 50 millions d'euros paraît élevé la proposition que nous faisons, c'est une demande de retrait au profit d'amendement numéro 91, porté par la commission des affaires pardon des je répondrai aux deux amendements identiques, qui sont le 87 et le 185 portées par monsieur barbarie et Monsieur Salmon

excusez-moi pardon lors de l'audition et je dois aussi dire que s'Nada, depuis 2011 qui me tient à coeur parce que je me suis battu depuis 11 ans sur le maintien de ce fonds et donc je tiens à remercier, je salue le la porte ouverte que monsieur le ministre a fait dans le cas du Fonds Vert et donc, en tout cas à titre de la commission des finances ces deux amendements il y a un avis défavorable, mais évidemment à titre personnel, je suis favorable. le deux le deux cent hausse des crédits du programme plan France très haut débit en faveur du déploiement du réseau à Mayotte, le déploiement du réseau haut débit à Mayotte connaît un un retard certain, nous le savons, un nouvel appel à projets, réseaux d'initiative publique sera lancée, selon le gouvernement, en 2023 à Mayotte, mais avec des crédits limité, or il est nécessaire de mettre en oeuvre des moyens plus conséquents au service de l'égalité nos territoires, c'est donc un avis favorable. pour la commission des affaires économiques, c'est le même amendement qui a simplement c'est le gage qui diffère. Donc c'est un amendement qui propose monsieur Guy et une hausse de de 20 millions d'euros, des moyens de la de la DGCCRF. Nous comprenons bien le sens de votre amendement dans un rapport de contrôle portant sur la DGCCRF adopté par la commission des finances en septembre dernier, nous avons d'ailleurs souligné les limites de la forte baisse depuis 15 ans, des moyens de la DGCCRF, en particulier d'un point de vue humain. Nous avons ainsi préconisé d'établir un effectif socle de cet agent par département, par le biais d'une légère hausse des effectifs. Dans un rapport de juin 2022 sur l'information du consommateur, la commission des affaires économiques, il avait d'ailleurs évoqué ce sujet. Néanmoins il faut noter que le PLF pour 2023 va dans le bon sens,

d'autre part, les crédits de la DGCCRF augmente légèrement de 2 5 % on a eux, ce qui représente 6 virgule 1 millions d'euros et 3 1 en crédits de paiement, ce qui représente 7,5 millions d'euros. Il ne nous semble donc pas nécessaire d'augmenter les crédits de la DGCCRF pour 2023 nous serons toutefois je me tourne vers Monsieur le Ministre, très vigilant quant à l'exécution des crédits et des emplois.

Ensuite, l'amendement 196 territoires d'outre-mer, la continuité territoriale doit en effet également le service postal sur le principe, nous sommes d'accord avec votre amendement qui vise à rehausser la dotation du groupe La Poste, pour permettre d'assurer une réduction de l'écart de prix de l'envoi des lettres et colis depuis et vers l'outre-mer en revanche angle budgétaire ne répond pas forcément aux enjeux que vous soulevez coup de dédouanement TVA octroi de mer pour ces raisons, nous ah mais nous émettons, pardon, un avis de sagesse et invitant le gouvernement à répondre globalement à cet enjeu. Il reste maintenant 188 monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président, donc c'est l'amendement présenté par Monsieur Barry, qui vise à une augmentation. 3 millions d'euros des crédits du programme 134 pour créer un chèque pour la transmission d'entreprise, la transmission d'entreprise est un enjeu majeur pour l'économie de notre pays, cet amendement, qui est issu de la délégation aux entreprises propose une solution intéressante en créant à financement pour limiter les coûts liés à la transmission d'entreprise. Néanmoins, il nous semble important de déterminer avec précision ses modalités et les clauses anti-abus, donc c'est une demande de retrait.

à l'occasion de notre mission de contrôle sur la DGCCRF, nous avons constaté la baisse des subventions en faveur des associations de consommateurs. Selon les informations que nous avions recueilli en 2011 4 38 millions d'euros étaient versés aux associations de consommateurs contre 2,25 millions en 2021. Soit une baisse de près de 50 % en 10 ans, néanmoins nous considérons aujourd'hui que le nombre d'associations de consommateurs doit être réexaminée, notamment par rapport à leur nombre, il nous semble important dans dans un 1er temps de mener une réflexion sur l'organisation globale avant d'augmenter les crédits et donc la proposition, c'est ta retraite. Et maintenant, il faut faire la même revue pour l'avis du gouvernement, mais c'est pas, c'est

près de 2 milliards d'euros de crédit pour les entreprises de la filière événementielle, on ne s'est pas arrêté là, évidemment, et dans le cadre du plan de relance, et même après le plan de relance, nous avons mis en place un un plan sectoriel dédiée de 100 millions d'euros et Jean-Baptiste Lemoyne, qui est là, le sait bien puisqu'il a porté, évidemment, ces mesures importantes qui permettent de garantir une mobilisation de presse sur fonds d'épargne pas la banque des territoires pour financer des projets de long terme de monter en qualité de la filière événementielle il ne ne nous semble pas nécessaire d'abonder de 500 millions d'euros

puisque, on met en place de évidemment de nombreuses actions d'ores et déjà, pour maintenir l'activité économique, on a eu l'occasion d'en discuter de manière très dense et très nourrie sur le PLF dans un contexte de crise énergétique, notamment en cas de rupture d'approvisionnement énergétique temporaire, on a une cellule d'anticipation qui nous permet passerait en cas et ce qui se passera en cas de rupture d'électricité sur le gars, je rappelle que nos stocks de gaz sont remplis à 99 % sur l'électricité, le dernier rapport de RTE a indiqué qu'il n'y avait pas a priori de risques de coupures au mois de novembre et décembre qu'il peut y avoir un risque en janvier selon évidemment la température et l'activité on s'y prépare, on anticipe des scénarios, y compris de délestage il y a pas lieu de penser qu'ils seront activés aujourd'hui, mais vraiment tout est fait en oeuvre tout est mis en oeuvre pour anticiper cela et être au soutien des entreprises avec les dispositifs nécessaires, je crois que le 192 c'était le même donc défavorable également, je passe au 89 de monsieur Montaugé sur territoire d'industrie défavorable également, moi, je veux rappeler que c'est un programme et vous l'avez fait d'ailleurs qui est saluée par unanimement voilà par les élus, les industriels, qui a apporté des résultats je crois probant pour la réindustrialisation nos territoires avec 2400 projets qui ont été financés, on a annoncé un prolongement de ce programme pour la période 2023 2026 en le concentrant sur 4 grands axes stratégiques que je ne me rappelle pas la définition de la future offre de service du programme, en lien avec les opérateurs partenaires est en cours, mais l'offre n'étant pas encore précisément arrêtée l'allocation de moyens supplémentaires financiers comme le propose le présent amendement n'est pas pertinente, néanmoins, compte tenu de l'enjeu et des soutiens du programme une discussion approfondie sur les moyens dédiés au programme et réunissant toutes les parties prenantes se poursuit, je passe au 207 de madame bla Trix compta, c'est également un avis défavorable sur les moyens d'action de l'agence Business France il y a, je l'ai rappelé dans mon intervention liminaire des moyens importants qui sont mis, il y a un point que vous avez évoqués sur la comparaison avec d'autres agences européennes, moi, je veux rappeler que Business France outre la subvention publique, et le chiffre d'affaires liées à son activité perçoit également des revenus en lien avec sagesse, sa gestion du dispositif VIE et enfin, je veux rappeler que le dispositif du chèque relance Export était destinée à répondre à un besoin conjoncturel lié à la crise et non à opérer un soutien structurel à des entreprises exportatrices il s'achève donc en fin d'année après un grand succès, près de 16000 chèques attribué pour 27 millions d'euros,

qui est pas tout à fait le même fonctionnement mais qui répond à des objectifs comparables les calibrage des critères et l'organisation de cette enveloppe est en cours par mes collègues du ministère de la transition écologique et je pense que la discussion de la partie de et du Fonds Vert vous permettra d'obtenir des garanties sur ce sujet-là, l'amendement numéro 200 de monsieur chaises sur Mayotte, je donne un avis défavorable, parce qu'il me semble satisfait puisque 4 à 5 millions d'euros sont prévus en PLF 2023 pour permettre le financement du projet il y a eu, je crois en 2014, 2015, un chiffre qui avait été évoqué effectivement de 22 millions de 27 millions d'euros, mais en fait, vous savez que l'intégralité des projets et des enveloppes ont été revus à la baisse, ensuite et le chiffre du du du financement anticipée du projet pour Mayotte, c'était quatre millions cinq effectivement il y a eu je crois un loupé dans le cadre du plan de relance ou l'enveloppe prévue n'a pas été fléché au bon endroit, mais on prévoit en PLF 2023 4 millions cinq précisément pour ce projet mahorais et donc là en tout cas l'intention me semble satisfaite, de monsieur Guey défavorable, j'ai indiqué les moyens. Supplémentaires qui étaient accordées à la DGCCRF ne semble pas nécessaire ni possible d'aller plus loin, comme le propose votre amendement mais il nous permet de redire tout notre soutien aux agents de cette très grande et belle direction l'amendement numéro 88 de monsieur babary, toujours sur la DGCCRF même avis pour les mêmes raisons défavorable, l'amendement de Madame Jasmin sur La Poste, on a eu l'occasion d'avoir le débat en PLF il y a des amendements qui étaient déposées, je crois que vous étiez là il y a l'activité dédouanement qui est maintenant confiée à à la Poste, c'est la conséquence d'une directive européenne, on ne peut pas s'y dérober, on n'a pas le droit en matière de droit européen de financer ou de compenser cette action à la Poste, c'est ça serait illégale du point de vue du droit européen pour être condamné pour cela, la France, en revanche, on a bien le problème très préoccupé par ce problème et on on a bien à coeur d'y répondre, mon collègue Carenco s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet, on travaille, on discute avec La Poste, pour qu'elle revoie notamment ses tarifs, il y a notamment le sujet des colis d'envoi non commerciaux avec la fameuse franchise à 200 euros

de 400 on reporte un peu le problème nous ce qu'on veut, c'est faire baisser les tarifs et on y travaille avec la Poste mais je sais bien que tant qu'on n'aura pas de résultat, il n'y aura pas de satisfaction, c'est normal, vous nous attendez sur ce sujet là, mais on va continuer à avancer, l'amendement 188 de Monsieur Babary toujours et toujours un avis défavorable sur le sujet. Lancement d'un chèque pour la transmission d'entreprise, on a des dispositifs fiscaux majeur pour la transmission d'entreprise, on en a parlé en partie hein de ce de moi, je veux rappeler le pacte Dutreil je vais rappeler l'exonération de plus-values de cession pour des entreprises individuelles, je veux rappeler les déclinaisons de tout ça en matière agricole, on a d'ailleurs retenu un amendement sur le sujet à l'Assemblée nationale, qui se traduit dans le texte, donc le le dispositif que vous proposez ne semble pas utile pour ces raisons-là et enfin nous arrivons sur l'amendement, c'est bien le dernier le 194 de madame bla Trix sur les associations de consommateurs et je veux bien ma petite note sur le sujet, merci. Les frites intéressant, on a besoin des associations de de consommateurs évidemment il mène une action, elle mène une action qui absolument essentiel dans le cas de la protection des consommateurs pour les informer, pour les accompagner dans les litiges qui qui peuvent les opposer aux professionnels conscients de la nécessité de cette action et les efforts réalisés ces dernières années, nous avons fait le choix d'inscrire dans le PLF un montant de crédit de 5 1000000 880000 stables par rapport aux exercices 21 22 qui permettra aux associations de remplir leur mission au vu de la densité du mouvement consumériste, il n'est pas possible d'augmenter les crédits qui lui sont alloués sans engager une réflexion approfondie sur sa structure. Dans ces conditions, c'est un avis défavorable, j'ai donné que des avis défavorables mais je ai précisé que dans la série suivante je donne quand même 2 avis défavorables, 2 avis

donc sur le 191 à retrait de la commission avis défavorable du gouvernement, c'est là que j'ai une demande de d'explication de Monsieur Lemoine, qui a la parole. soumis cette proposition à à notre assemblée dans en tous les cas pour ouvrir le débat pour qu'on ait l'occasion je crois de signaler au gouvernement tout l'attachement qu'on a au fait de de soutenir le secteur événementiel parce que ils participent à la vitalité de nos territoires, les foires, les salons, les congrès et etc, on s'est sont sont très importants et la mécanique qui est proposé, alors c'est une masse financière 500 millions d'euros, mais en lisant exposé des motifs, je trouve les mécaniques très intéressante parce que justement le rapporteur évoquait le droit européen et les limites qu'il peut mettre en en termes d'aide mais justement on ne serait pas sur un système d'aide on serait pas sur un un système de de subventions, on serait sur le fait que ces entreprises les ETI qui sont leaders dans, dans, dans le secteur dans le monde, émettre des obligations convertibles en actions à échéance 10 ans par exemple, et ça, ça s'assimiler à des quasi-fonds propres et donc ça aidera le secteur effectivement à repartir à investir et donc voilà le le message envoyé au gouvernement, c'est que, on souhaite qu'ils puissent travailler à ce type de dispositif, hein, mais voilà, je pense que c'était un amendement d'appel et merci de l'avoir soulevé.

j'aimerais être autant optimiste que vous sur le risque de délestage, je ne le suis pas autant, mais j'espère que vous aurez raison et que nos entreprises n'auront pas à utiliser leur groupe électrogène qui fonctionne au fioul parce alors là pour avoir voulu arrêter le nucléaire, ce serait vraiment pire que tout.

Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais effectivement appuyer la démarche présentée par notre collègue dans dans cet amendement par rapport aux territoires d'industrie parce que Monsieur le ministre, il y a une relative urgence, on est à l'échéance des crédits d'ingénierie et aujourd'hui on ne sait pas de quel moyen les territoires vont disposer au 1er janvier 2023 pour poursuivre effectivement la démarche des territoires d'industrie dans le cadre du plan d'investissement France 2030 sur lequel effectivement il y a des enjeux importants pour les territoires et l'état peut pas à la fois promouvoir ce dispositif et ses engagements et ses orientations et ne pas donner aux territoires les moyens d'ingénierie pour leur permettre de les mettre en oeuvre, en particulier dans les territoires les plus ruraux sur lesquels l'industrie et présente, je pense en particulier au bassin qui qui qui touche le Cantal, l'Aveyron et le et le l'autre qui est aujourd'hui autour de la mécanique vallée du bassin industriel du d'Aurillac à un territoire d'industrie qui fonctionne bien et qui est en plein d'interrogations quant à son avenir au regard des manque du manque des crédits d'ingénierie, je vous remercie. Donc je mais on voit ses rendements 89, sagesse, la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Quels sont ceux qui sont contre. Il y en a pas abstention cet amendement là et donc adopté, nous passons 207 avec Éric de retrait de la commission défavorable du gouvernement

D'accord, donc il a été retiré, non, il y a pas été retiré, donc je préfère qu'on fasse le vote pour que personne ne soit frustré, donc qui est pour l'amendement 207.

pas l'abstention n'est pas adopté. Le 87 ensuite, avec avis défavorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour, Désolé, je ne veux pas prolonger les, les, les débats mais je je je me je suis quand même un petit peu interrogatifs pour avoir participé à tous les débats ou presque depuis la première partie, on a encore entendu Monsieur le Ministre, mettre en avant le fond Vert et j'ai un peu de mal à voir le lien entre un rétablissement du Fisac ou ou en tout cas une action qui viendrait accompagner nos commerces proches du Fisac et le Fonds Vert, même si toutes et développement durable mais mais néanmoins je je ne vois pas bien le lien voilà je vous remercie.

L'abstention et donc adopté

avec passion ah ah et et connaissances et compétences c'est bien rappelé rappelé que reporter à la prise l'aide du plan France très haut débit pour les Mahorais serait considérablement inférieur aux autres territoires ultramarins et dont l'objet de cet amendement, il y a un tableau qui indique que la pour la Guadeloupe 350 euros par prise subventions la Guyane 772 la réunion

tout en regrettant, votre vie, Monsieur le Ministre défavorable. Entendu donc sur cet amendement Monsieur le Lemoine rajouter un mot. le gouvernement était défavorable, mais parce qu'il considérait que les moyens étaient là, d'une façon d'une autre, donc on comprend qu'il y a, il y a, il y a une adhésion en tous les cas à l'idée de pouvoir accélérer ce déploiement, ce qui est sûr, c'est que, effectivement, les collègues locaux ont travaillé, je veux, je veux dire combien le sénateur Thani Mohamed Soilihi également être attaché à la mise en oeuvre de ce programme et que pour cette raison, voilà, nous allons également le le voter en en pensant que,

tout le monde donc à travers le plan cuivre France Télécom de l'époque et et ils ont pas ils ont pas les supports alors que il n'y a que 18000 lui lignes en cuivre pour 50000 logements, donc on ne peut pas prendre appui sur les supports de de du cuivre pour pouvoir développer la fibre d'où la nécessité des 22 1000000 Donc je peux mettre aux voix cet amendement 200 avec donc un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, abstention, il est donc adopté ensuite de 200, avez un avis de retrait, madame la présidente. Pardon, Monsieur le Ministre, je voudrais juste rappeler à nos collègues qui reste presque vingt minutes il nous reste quelques amendements et ça serait bien qu'on soit concis dans l'expression voilà si je peux me permettre ce conseil merci et qu'on termine à une heure et demie merci beaucoup.

prenons l'exemple vingt sont volontaires, les quarante reste seront qui-t-il considéré en sur, effectif et sera-t-il une incidence sur évidemment le recrutement de septembre 2023, mais je me permettrai de vous poser ces questions par écrit, je vous remercie et je remercie monsieur le rapporteur de son avis favorable personnel. Entendu donc. Sur le 200 hein, j'ai un avis de retrait si j'ai un avis de retrait de la commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

abstention il est pas adopté. Nous avons encore le avis de retrait de la commission avis défavorable du gouvernement. Monsieur une Paris. Juste un mot pour considérer que ce que j'ai donné comme exemple notre collègue Fabien, c'est-à-dire 20 emplois qui seraient transférés soixante qui seraient conservés, c'est pas qu'un exemple, c'est la réalité, et donc c'est 60 postes, ils vont être décompté dans la capacité de la DGCCRF d'embaucher, or je rappelle que chaque année il y a 145 départ dans l'ensemble de la DGCCRF et pour cette raison, je maintiens mon amendement. Entendu donc qui est favorable à cet amendement 88. Avis contraire. Abstention : il est adopté, Besancenot 196 avec un avis de retrait de la commission, un avis défavorable du gouvernement Madame Jasmin. Vous demandez à parole. J'ai pas entendu au retrait, j'ai entendu sagesse et. S'il s'agissait de la commission sagesse de la commission oui alors, oui, oui, exact. en même temps je voudrais justement, Monsieur le Ministre, j'ai entendu vos arguments, mais la Poste et financée par l'État et le fonds de péréquation abondé pour couvrir en partie s'est c'est une solution qui permettrait justement d'assurer cette continuité territoriale et et d'éviter justement les complications qui casse la tête de Monsieur le Ministre délégué parce que lui il sait pas comment faire, il me l'a dit, il m'a dit c'est complexe, mais là c'est une possibilité qui ne pourrait pas pas gêné en quelque sorte avec les arguments que vous avez donc en tout cas, chers collègues, je vous demande le soutien parce que ça ne va pas forcément, c'est une des solutions possibles. Je me vois cet amendement, qui est pour.

Non, monsieur le Président, je vais maintenir cet amendement parce que j'ai bien entendu les propos du mini sur les aides qui sont déjà apporté pour la transmission mais le pacte Dutreil ne correspond pas du tout, au type d'entreprise que j'ai cité, il s'agit des TPE et des toutes petites PME par connaît bien le pacte Dutreil qui s'adresse à des entreprises qui transmettent d'une façon familiale, l'entreprise c'est pas du tout le cas et on cherche désespérément à la délégation aux entreprises, le moyen d'aider et d'anticiper, surtout pour les chefs d'entreprise leur départ. Donc cet amendement 188 et maintenu, quels sont ceux qui sont pour.

194 de madame la triple compta avec avis de retrait. De la commission et avis défavorable du gouvernement. Il est maintenu, donc je mets aux voix qui pour.

ce sont des emplois de qualité non délocalisables qui fabrique du lien social et de la qualité de vie, l'ESS concerne en tout de 7 millions d'employes dans plus de 60 % de femmes dans plus de 200000 entreprises pourtant les moyens dédiés à l'action, numéro 4 du programme 305 Stratégie économique reste stable cette année, marquant ainsi un recul relatif, alors que le budget de la mission augmente sensiblement, c'est pourquoi cet amendement propose de renforcer les moyens de l'ESS de 20 millions supplémentaires, je vous remercie. Oui, monsieur le président, donc sur l'augmentation de 20 millions d'euros des crédits, donc de l'action et l'économie sociale et solidaire, responsable sur le programme 305 l'économie sociale et solidaire et la fauteuil un secteur déjà un déjà un important de notre économie, un sujet d'avenir, l'augmentation des crédits que de vous proposer pour l'action du programme, sortir à Paris néanmoins élevée, elle représente une hausse d'environ 100 pour 100, donc c'est un avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement avec un double avis défavorable qui est pour. Attention, il n'est pas adopté le 90 Monsieur Montaugé. monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, dans le droit fil des, des, des travaux de la commission des affaires économiques qui ont été menées par la présidente Sophie Primas Amélie hacker et moi-même, des des formuler des préconisations pour améliorer la souveraineté économique nationale et parmi ces préconisations figurent la réalisation d'une cartographie permettant

quand on ne peut pas ne disposer voilà donc on propose d'affecter 12 millions et demi d'euros à la réalisation de cette cartographie et à l'élaboration d'une stratégie

mais. Merci monsieur le le président monsieur le ministre et chers collègues, il s'agit ici, alors il en a été beaucoup question au cours de la soirée, notamment dans le dans le débat général de renforcer les les moyens de de fonctionnement de de Business français voilà pour développer évidemment le chiffre à faire de nos entreprises françaises à à l'étranger à l'export dans un contexte, ça a été rappelé également de dégradation extrêmement forte de la balance du commerce et extérieur, voilà, avec un déficit qui est qui est au-dessus de 150 milliards d'euros Business se fait l'excellent : je rappelle le contexte d'inflation dans lequel on est qui est, qui est supérieur à 5 % donc on demande, on demande de 8 millions de mémoire, c'est 8 millions huit mille 8 millions d'euros de budget supplémentaire, bon ça fait à quelque chose de près en tenant compte de l'inflation ne maintiennent des moyens, mais les moyens qui sont, qui sont absolument nécessaires. Madame, monsieur, à votre avis. C'est un avis favorable. Monsieur le Ministre. Je mets aux voix cet amendement 91 avec avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Contre l'abstention, il est adopté sur la presse et notamment, il y avait une sagesse du gouvernement et ceux qui lève le voile. Sur l'amendement précédent qui a été voté avec une sagesse de votre part est-ce que vous levez le gage monsieur Ministre le

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent donc dans un but d'inciter les entreprises à convertir leurs groupes électrogènes fonctionnant au fioul en groupes électrogènes fonctionnant avec une énergie moins productrice de CO2 voilà incitation et accompagnement. La commission. C'était une proposition de retrait, c'est un sujet que nous avons évoqués précédemment. Je le retire, et je ne refais pas mes même remarque, mais voilà, elles sont toujours là. Merci madame comptable pour le 180 148. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, cet amendement a pour objet de, de, de mieux financer les crèches, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui sont un maillon essentiel de l'ESS la loi Hamon a confié au Crest de multiples missions défend des intérêts des entreprises de l'ESS apporter un soutien à la création développement maintien des entreprises soutenir la formation des dirigeants des ça des des salariés, et aujourd'hui on s'aperçoit que les crèches sont très clairement sous-financé, elles sont, c'est un rapport de l'Assemblée nationale qui l'indique 50 elles ont cinquante pour moins de ressources que les chambres de commerce et d'industrie ou que les chambres des métiers, donc il est vraiment utile pour développer l'ESS de mieux. Financer les crèches, c'est pour ça que nous proposons un financement supplémentaire de 1 virgule 5 millions d'euros.

le présent amendement a pour objet de rétablir l'action vingt afin d'affirmer la nécessité du financement budgétaire de l'activité de garantie de BPI France l'un des piliers de la politique publique de la transmission d'entreprise, attendu en France, la dotation et pour l'année 2023 symbolique 10000 euros car le financement est assuré via les crédits du plan de relance la dotation devrait être bien plus conséquente en 2024 année pour laquelle le financement des activités de garantie ne sera plus assurée, le risque étant la diminution des aides de BPIFrance pour soutenir les reprises de TPE et PME présent amendement a donc pour objectif de faire acter le principe du rétablissement de la ligne de crédit dédiés à se dire. Positif.

Oui : avis défavorable, même si on travaille évidemment avec les pays France sur son prochain plan d'orientation stratégique et les différentes missions qui devront être financés. Je mets aux voix l'amendement avec favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Et contre. Censure il est adopté, nous allons pouvoir voter sur les crédits de la mission Économie figurant à l'état B il n'y a pas eu de demande d'explication de vote je rappelle pas la commission des finances, est favorable à l'adoption de ces crédits, je mets aux voix la mission qui est pour. Contre. C'est accepter, il faut appeler en discussion, l'article 43 qui est rattaché à crédit, la mission de il faut que nous nous prononcions sur l'article 43, qui est pour. pour. Il est adopté, après l'article 43, nous avons un amendement présenté par le rapporteur de la commission des finances. Oui, monsieur le président, merci le présent amendement vise donc à prolonger d'un an, le dispositif de prêts participatifs pour les petites entreprises et positif qui a été mis en place à l'initiative du Sénat en 2020 lors de la Cristiani, terre, il a été déjà plusieurs fois prolongée, notamment notre initiative à celle du rapporteur général l'amendement donc propose de prolonger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2023, tout comme le fait par ailleurs le présent projet de loi de finances pour le prix garanti par l'État, article 37 bis merci Oui c'est un avis défavorable, le dispositif a été prolongée à 3 reprises depuis son lancement et une nouvelle prolongation au-delà du 31 décembre 2022 ne nous semble pas opportune, on assiste en effet d'abord à une forte réduction du flux de nouvelles demandes mensuelles qui est passé de 150 en 2021 à 45 sur le 1er semestre 2022 depuis juin, plus aucune nouvelle demande n'a été formellement adressé, ça montre que le vivier d'entreprises éligibles au dispositif s'est tari ensuite le dispositif plafonnés à 100000 euros ne répond pas en tant que telle, aux conséquences du conflit en Ukraine, tandis que les aides spécifiques qui ont été mises en oeuvre pour ce qui concerne la hausse du coût de l'énergie, ils répondent enfin il faut rationaliser le nombre de dispositifs d'aide aux entreprises à des fins de clarté, de lisibilité.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, ce tu amendement porte sur une demande de rapport, je sais que le Sénat n'en est pas particulièrement friand, mais il me semble utile car il contribuera à faire le point sur les crédits mobilisés par l'État et par les collectivités pour le développement et le soutien de l'ESS en l'absence d'un document budgétaire et d'un CF SS, il est difficile de prendre la mesure des politiques publiques qui visent au qui impacte l'ESS et donc cet amendement permettrait de produire un rapport d'information complet complet facilitant le changement d'échelle de l'ESS. économie dont la résilience l'intérêt dans cette période pour la transition écologique pour la transition sociale et reconnu, je vous remercie. il s'agit de d'une demande de rapport sur l'intervention des personnes publiques en faveur d'économie sociale et solidaire, c'est un sujet effectivement très important mais on on se dit qu'un document budgétaire serait peut-être plus approprié et donc c'est une proposition d'une demande de retrait.

Le ministre de raccourcis pas le délai le le débat, bon je mets aux voix cet amendement donc avec avis favorable du gouvernement et la de retrait de la commission qui est pour. Alors il y a des pour.

nous en parlerons nous allons encore avoir un amendement sur les prêts et avances à des particuliers, l'état des amendements de nos rapporteurs, le numéro 14 messieurs Cosic. Et merci Monsieur le Président, donc : le programme 868 pré-avance pour le développement du commerce avec l'Iran, a été créé par la loi de finances pour 2018 au sein du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, l'objectif de ce programme était de permettre à l'État d'accorder des prêts à BPIFrance pour financer le dispositif que BPI France était en train de mettre en place pour soutenir les entreprises françaises souhaitant exporter leurs produits en Iran, la loi de finances pour 2018 avait ainsi autorisé le déblocage d'un prêt de 100 millions d'euros en autorisations d'engagement toutefois l'entrée en vigueur de sanctions économiques américaines contre l'Iran à compter de novembre 2018 a conduit BPIFrance à suspendre le projet, son directeur général, estimant que les conditions n'étaient plus réunies pour le mettre en oeuvre en conséquence que programme 868 n'a pas connu de consommation de crédit depuis sa création, sa suppression doit dont être décidé après plusieurs années sans utilisation. Je me revois cet amendement, la commission de la commission avec avis favorable du gouvernement qui est pour. Entre l'abstention est adopté, nous allons voter sur le compte spécial Prêts et avances à des particuliers, organismes privés, pas de demande d'explications de vote, la commission est favorable, je mets aux voix le crédit pour. Entre adoptée et ben, écoutez, mes chers collègues, conformément au planning et au sommet de la présidence, nous avons terminé à l'heure je vais lever prochaine séance vendredi 25 à 10 heures 30 pour la conclusion, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le PLFR 2022, la séance est levée.